est reprise avec une mise au point de Madame Jourda sur un vote. Merci madame le président pour. Faire la mise au point effectivement suivante sur le scrutin public numéro 297, mes collègues Jacqueline Eustache-Brinio et Arnaud Bazin souhaitaient voter pour. Ah que vous en ai donné, madame la sénatrice, elle sera transcrite au Journal officiel et nous reprenons la discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice, 2023 2027. Nous sommes parvenus à l'article 21. Et nous commençons par un amendement de monsieur le garde des Sceaux 273. merci madame la présidente. Il s'agit par cet amendement de rétablir. L'article 21 prévoyant une prolongation du délai d'habilitation. À réformer le droit de la publicité foncière. Alors cet amendement. Donc je viens de le dire, a pour objet de rétablir l'article 21 qui a été supprimé en commission. Les premiers travaux menés ont révélé en réalité que l'élaboration de la réforme de la publicité foncière. Nécessite un travail inter-ministériel conséquent. Pour obtenir un résultat cohérent entre la partie législative et la partie réglementaire. Deuxièmement, un temps d'échange et de consultation suffisant avec les parties prenantes ces différentes phases d'élaboration du texte requièrent encore plusieurs mois de travail. Et le gouvernement voulant. Conduire à son terme cette réforme. Tant le ministère des Finances et le ministère de la justice souhaite rétablir la prolongation de l'habilitation. Réforme a reformé pardonnez-moi le droit de la publicité foncière. Quel est l'avis de la commission. Madame la présidente. L'avis de la commission sera défavorable en effet. Vous aviez déjà 18 mois pour le faire. Le problème de ces habilitations et vous savez bien que nous n'aimons pas les habilitations, c'est que pendant ce temps là. Le Parlement abandonne sa compétence et sur un sujet majeur. Donc ça ferait presque trois ans. En tout, les 18 premiers mois et des mois suivants, que vous ne Donc. Bah pendant la navette si vous raccourci scié peut être qu'on pourrait regarder les choses. Parce qu'on comprend que ça se termine au mois d'août et que ça peut être compliqué de finir au mois d'août mais entre ne pas finir au mois d'août. Et redemander 18 mois il y a probablement. Il y a un moyen terme. Donc pour l'instant c'est défavorable mais si vous voulez métier par exemple à la fin d'année 2023. Peut-être que cela peut être entendable en tout cas défavorable pour l'instant. Monsieur le Ministre. Je vois ça avec Bercy au plus vite et je vous propose de raccourcir. Oui. Mais c'est une rectification. C'est-à-dire que. Je vais mettre au vote cet amendement là il est vous le rectifiez, Monsieur le Ministre, Non très bien. Donc je mets au vote ainsi avec un avis défavorable de la commission qui est pour l'amendement du gouvernement. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'article 21 et donc supprimer nous passons l'article 22 avec un amendement toujours du gouvernement l'de 175. Merci madame la présidente. Cet amendement modifie les conditions statutaires. Permettant le passage au grade de premier conseiller pour le coeur des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Avis de la commission. Ce sera un avis défavorable. Madame la présidente, parce que nous n'avons pas eu le temps de mener les auditions pour comprendre les effets de cette mesure. Donc pareil à ce moment du débat, je pense que il vaut mieux rester un avis défavorable. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est pour.

Qui est contre. Qui s'abstient il était adopté après l'article 22 l'amendement 153 monsieur Bena Roche. Merci madame la présidente. Cet amendement de des pas supplémentaires de vice-président que ça des tribunaux administratifs. Donc il est clair que. On a mis en évidence souvent y compris dans le cadre de de de l'étude de cette loi, l'abondance des contentieux. Les interminables délais de procédure, la charge de travail exponentielle des professionnels de la justice et que tout cela nécessite de déployer des moyens supplémentaires dans la création d'emplois, on le sait, on en a parlé et certains ont été affectés et nous saluant une nouvelle fois les efforts fournis entre autres en 2016 quand il avait eu la création de postes additionnels de 1er vice-président dans les tribunaux administratifs qui sera composé de 8 chambres ou de plus de 8 chambres. Néanmoins, si cette initiative souligne la préoccupation du gouvernement sur cette question. Ces avancées ne masque pas des difficultés qui sont persistantes et donc nous sommes pour une persistance aussi dans les efforts. Que nous encourageant pour l'instant mais. Que nous encourageons, être encore plus important. Dans le rapport sur le projet de loi de finances 2023. Je suis c'est c'est dans ma mission, donc je suis rapporteur de ce budget pour le. Pour le Sénat au nom de la commission des Lois, il est précisé que le niveau des affaires reçues dans les tribunaux administratifs en 2021 dépassé de près de 4 5 % celui déjà exceptionnellement élevé de l'année 2019. Nous proposons donc levier puisque c'est le terme utilisé pour des tas de raisons actuellement. Supplémentaire pour sortir de cette situation inquiétante, en demandant la création systématique de poste de vice-président pour les tribunaux d'au moins 5 chambres, les tribunaux administratifs composé d'au moins 5 sobre. En raison du sous-effectif criant certains syndicats espèrent même la possibilité de poste de vice-président dans des tribunaux administratifs à deux chambres dès que la charge de travail, l'organisation de ce dernier le nécessite. En faisant cela nous permettra une justice plus fuite du sommet des juridictions jusqu'aux justiciables nos professionnels justice souffrent de ce sous-effectif épuisement des missions dépression et cetera. Nos magistrats, greffiers, président vice-président se noie dans le renforcement des contrôles, je le ferai en explications. Quel est l'avis de la commission. néanmoins sans surprise comme c'est une demande de rapport nous émettrons un avis défavorable. Il y a une façon de réparer cela c'est de voter le texte mardi. Très bien je vais donc mettre aux voix c'est monsieur Ménard Roche pour une explication de vote. Sur certains points, nous aurions sûrement mon pour l'sûrement voter ce texte là on en décidera mardi. En fonction d'un certain nombre d'éléments négatifs qui sont restés voire même qui ont été amplifiées. Dans ce texte. Après coup, pour, pour terminer sur le sujet qui était celui de la justice administrative. En dehors de cette création. Alors on a demandé un rapport, parce qu'on n'a pas la possibilité bien entendu nous même de demander la création de de de de ces postes là puisque ça serait une recevabilité. C'est pour ça qu'on demande un rapport si les décisions ont été prises de les créée par le ministère ou que le gouvernement faisait de lui-même un amendement pour les créer ça nous irait aussi parfaitement bien juste pour dire qu'il y a une autre demande alors qui qui a été déclarée recevable là aussi parce qu'elle crée des des pas supplémentaires mais que de vous, vous devez connaître d'un certain nombre de magistrats c'est la possibilité de prêter serment et de porter la robe. Donc je je me fais je vous fais part de cette de mode, vous connaissez en dehors de tout amendement. Bien je vais mettre aux voix cet amendement. 153 qui a reçu un avis défavorable de la commission un avis de sagesse du gouvernement qui est pour. Qui est pour. Qui est content. Il n'est pas adopté. Si madame la présidente, j'ai l'honneur de porter de présenter cet amendement qui est porté par le Conseil d'État. Il a pour objet de rétablir la mesure qui intègre les nominations de conseiller référendaire en détachement dans le calcul du nombre de nominations de conseiller mettre au tour extérieur. il est pas obligée également. De rétablir la mesure de raccourcissement de la durée des fonctions de président et de vice-, présidents de chambre régionale des comptes. La réforme de la fonction publique. Amorcée depuis maintenant 2 ans. A profondément rénové les parcours de carrière et d'encadrement supérieur de l'État. L'ordonnance du 2 juin 2021. Ainsi modifier les principes de carrière des magistrats de la Cour de comptes et des magistrats des Chambres régionales des comptes, la déclinaison au niveau réglementaire des principes de carrière et de rémunération de l'encadrement supérieur est actuellement en cours de discussion devant le Conseil d'État. Sa mise en oeuvre impose de modifier les articles L 122 tiré trois L 221 tiré de du code des juridictions financières afin de donner sa pleine portée à ses nouveaux principes. D'une part la diminution du nombre de domination au tour extérieur des conseillers maîtres. Impose de rétablir le vrai sens donner à ces nominations en mettant fin à la distinction entre magistrats en activité et magistrat en détachement dans le calcul des promotions possible. Il ne faut pas non plus faire dépendre le nombre de ces nominations des choix de carrière des magistrats au moment de leur promotion. D'autre part et enfin la durée excessive des fonctions de président et de vice-, président de la chambre régionale des comptes de leur permettre de dérouler une carrière suffisamment diversifiée, en occupant au moins 2 postes successifs dans les mêmes fonctions. La mobilité sur ces postes stratégiques au coeur des principes de la réforme s'en trouvera accrue de magistrats un plus grand nombre de magistrats d'accéder à ces fonctions. Ce sera un avis défavorable. Madame la présidente, puisque l'amendement du gouvernement tend à rétablir le texte qui avait été modifié en commission des lois du Sénat. Concernant donc les juridictions administratives. Pourquoi nous avions supprimé de mesures qui ne nous paraissait pas justifié. Même si le Conseil d'État semble les porter d'abord pour une question de l'harmonisation des durées de fonction de chef de juridiction. Qui est de 7 ans aujourd'hui dans les juridictions judiciaires, donc on va harmoniser avec les juridictions administratives, ça nous paraît cohérent ensuite. Effectivement l'ordonnance de 2021 concernant la haute fonction publique d'État a beaucoup à modifier les parcours et les carrières. Néanmoins, il me paraît un peu. Prématuré aujourd'hui d'en avoir les effets de pouvoir la modifier à nouveau, toujours dans ce souhait de de stabilité que nous portons et enfin dernière chose, vous nous dites que il y a encore un certain nombre de sujets qui sont en négociation et qu'il faut anticiper les résultats de ces négociations pour permettre leur application. Ça nous paraît être une méthode un peu étonnante. Bien je vais mettre aux voix cet amendement du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est pour.

il est adopté l'article 25 même vote il est adopté à l'article 26. L'amendement 27 qui est présenté par Madame de La Gontrie. Merci madame la présidente. C'est un amendement. Proposé par notre collègue Michel Meunier. Et qui souhaite. Supprimer. La disposition qui prévoit de transférer le juridique les les les le contentieux des juridictions de la tarification sanitaire et sociale. Vers les juridictions administratives de droit commun. On sait que ce sont des juridictions parent pauvre. Et. La question étant que de transférer ses compétences va amener une perte importante de la connaissance de ses sujets de l'efficacité donc de ce contentieux et donc de fait. Poser problème sur la qualité. De l'accompagnement De l'accompagnement des personnes vulnérables, protection de l'enfance, perte d'autonomie exclusion sociale ou maladie chronique, donc. Transféré pour rationaliser peut-être mais perdent de la compétence au préjudice du justiciable. C'est problématique donc nous proposons la suppression de cet article. Quel est l'avis de la commission. Sera un avis défavorable. Alors la commission des lois. A déjà préféré plutôt que de recourir à une habilitation d'inscrire dans le dur. Ce transfert de compétence. Des tribunaux intérêt j'régionaux pardon qui juge le contentieux de la tarification sanitaire et sociale. Parce que le rapport de la mission permanente d'inspection des juridictions initiative a mis à jour en 2020, un certain nombre de difficultés rencontrées par ces juridictions spécialisées dont le contentieux s'amenuise au fur et à mesure ces difficultés des relatives notamment à des questions de procédure et et. Aux règles de droit qui prenait de plus en plus de pas place dans ce contentieux, d'où l'importance de. De supprimer l'existence de ces juridictions pour que ce soit traité par les juridictions administratives de droit commun. Voilà et donc c'est pour ça que nous menons un avis défavorable de suppression. Monsieur le Ministre qu'est l'avis du gouvernement. Défavorable une précision supplémentaire que je souhaitais porter le volume du contentieux de la tarification sanitaire et sociale ne cesse de décroître de décroître depuis 2014. C'est un peu moins de 200 affaires qui sont traités par an en première instance et moins de 50 ans. Appel. Se voit cet amendement qui a reçu un double avis défavorable qui est pour.

même vote, nous passons à l'article 27 Monsieur Mohamed Saïdi. Vous avez la parole pour votre amendement 227. Oui madame la présidente. Cet amendement prévoit. La suppression de l'article 900 du code de procédure pénale. Qui adapte. Au plus beau département de France, je parle du département de Mayotte. L'article 706 tiret 14 relatif à l'indemnisation sous condition de ressources de certaines victimes d'infractions. L'article 900 n'est plus nécessaire dans la mesure où l'article 706 14. Il est pleinement. Applicable, sans besoin d'adaptation supplémentaire.

Un moment de coordination. Favorable, favorable donc pas d'avis défavorable dans l'hémicycle. Il est donc adopté et je mets aux voix l'article 27 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté à l'article 28, un amendement 285 des rapporteurs coordination. Monsieur le Ministre, car ça n'y voit d'inconvénient, il est adopté, je on voit l'article 28 qui est pour qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Un autre amendement de coordination. Le 286 des rapporteurs, monsieur le ministre, il vous convient. il ne heurte personne. Il est donc adopté le 28 là nous passons la parole à Madame de La Gontrie. Il tombe. Si madame de La Gontrie dit. vous confirmez. Il est retiré. On va dire. Bonsoir. Oui mais nous on va dire qu'il est retiré. je me vois l'article 29 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Nous en avons donc terminer avec l'examen des articles de ce texte. Je vous rappelle que les explications de vote et le vote par scrutin public. Auront lieu mardi 13 juin à 14h 30 et nous prenons maintenant. L'examen du projet de loi organique relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire. Je vous laisse 3 minutes pour fermer vos dossiers. Ouvrir le suivant. Changez. Les. Changer les équipes vendez commissaires.

mais c'était nous vous attendions et nous commençons avec un amendement 54. De madame la présidente Assassi. Oui merci madame la présidente, notre amendement visant à restreindre. L'autorité du. Garde des Sceaux, pas d'attaques personnelles bien évidemment à l'égard de de notre Ministre donc. Vise à restreindre l'autorité du garde des Sceaux à sa seule compétence en matière de politique pénale conformément à l'article 30 du code de procédure pénale qui énonce les attributions du du garde des Sceaux. Nous souhaitons donc souligner l'importance de maintenir une séparation claire entre les pouvoirs exécutif et judiciaire, selon l'article 30 du code de procédure pénale. Le garde des Sceaux est chargé de définir et de mettre en oeuvre la politique pénale de l'État. Cela comprend notamment l'élaboration des directives générales relatives à l'action publique et à l'exécution des peines, ainsi que la supervision des services pénitentiaires en limitant l'autorité du garde des Sceaux à la seule politique pénale notre amendement vise à préserver l'indépendance de l'autorité judiciaire, il s'agit de garantir que les décisions, les décisions judiciaires soient prises de manière indépendante sans ingérence ou influence politique. Nous continuons de défendre à défendre en laissant au pouvoir judiciaire, la responsabilité de prendre les décisions juridiques en toute ah partialité on renforce la confiance du public dans le système judiciaire enfin notre amendement est définitivement en adéquation avec les principes de séparation des pouvoirs et de l'état de droit en limitant le rôle du garde des Sceaux à la politique pénale on préserve nous semble-t-il l'équilibre entre les différents pouvoirs et on évite toute concentration excessive du pouvoir. Je vous remercie. Qui est de l'avis de la commission. Ce sera un avis défavorable. Madame la présidente, chers collègues, en effet, une telle disposition reviendrait à notre avis à réduire excessivement l'autorité du garde des Sceaux d'autant que le ministère public, dispose de compétences en matière non pénale comme l'état civil les nationalités et cetera donc il apparaît paradoxal que ses fonctions soient exclues par principe du Champ de l'autorité du garde des Sceaux, alors même qu'elles peuvent revêtir une sensibilité moindres que la matière pénale. Monsieur le Ministre. Merci madame la présidente. Madame. Madame la sénatrice. Il y a quelques jours. Jean-Jacques Urvoas ce mon prédécesseur a dit que le garde des Sceaux avait, au fond, peu de pouvoir. Et qu'il le déplorait. Alors évidemment il y a des sauts quelque pouvoir en ce qui concerne la politique pénale. Mais ses pouvoirs ne peuvent pas se réduire à cette seule matière, il y a. Là matière civile, commerciale l'enfance en danger. Et il y a de mon point de vue une nécessité absolue. D'avoir une politique unifiée et cohérente sur l'ensemble du territoire et une telle politique ne peut être défini et mené que par le gouvernement sur le contrôle du Parlement. Comme le rappelle d'ailleurs l'article 20 de notre constitution. Cette position a d'ailleurs été défendu par le comité des états généraux. Et je tiens à rappeler enfin que le Conseil constitutionnel. A jugé que cette autorité du garde des Sceaux sur les magistrats du parquet est conforme aux principes constitutionnels la suppression de l'autorité du garde des Sceaux dans ces domaines me paraît contraire à la Constitution et je le dis inopportune. Sur le fond je suis donc défavorable à cet amendement. Madame président. Oui. Merci madame la rapporteure. Merci monsieur le garde des Sceaux je je je je. Je pense que je vais retirer cet amendement parce qu'il me semble. À la lecture de la Défense que j'ai fait et puis de ce qui nous a été et dit que cela mériterait quand même un débat un petit peu plus approfondie que simplement. De de de de porter cette mesure par la voie d'un amendement dans un texte aussi important. Merci. Nous passons à l'amendement 38 monsieur Bonnecarrère. Indépendance et impartialité. De. Sujets importants au coeur de l'oeuvre de justice. Je crois qu'il n'y a aucun aucune interrogation sur le fait que ces 2 éléments sont consubstantiels de l'action d'un magistrat. Reste la question de l'action syndicale que nous nous remettons en cause ni de près ni de loin et dans lequel nous considérons tous syndicats et tout. Syndicats de magistrats également à une liberté totale d'expression cette liberté d'expression est parfaitement conforme aux logiques d'indépendance des magistrats. Reste la notion d'impartialité. Il nous semble que cette notion d'impartialité tellement importante que doit irriguer à la fois l'action personnelle d'un magistrat, mais qu'elle doit irriguer aussi l'action collective des magistrats en d'autres termes, nous ne voyons pas en quoi il pourrait y avoir une entrave à la liberté d'expression à l'expression collective des magistrats à travers la notion d'impartialité la notion d'impartialité c'est revient à ne pas porter atteinte à injustifiable ou à une catégorie de justiciables. Il me semble que l'on peut très bien porté, encore une fois la voix collective d'une profession et fortiori d'une profession aussi importante que celle des magistrats sans nous avoir une expression qui puisse mettre en cause une forme de partialité exprimé. Également, je crois que les magistrats ne peuvent pas douter de leur importance dans la société française de l'important c'est de la crédibilité qui doit être attachés à leur parole et qui et que tout ce qui s'explique toucherait dans une expression collective. À des éléments de partialité à mon avis elle affaiblirait la portée de cette voie. D'où l'amendement que nous présentons. Merci madame la présidente. Ce sera un avis favorable car nous pensons que cet amendement vient utilement rappeler que le droit syndical des magistrats doit être compatible avec l'impartialité qui est attachée au devoir de leur état.

que l'inscrire dans le. La loi n'est pas. Sans utilité. La commission a d'ailleurs précisé la définition de la faute disciplinaire et il y a inclus les manquements aux principes d'impartialité au sein de cette définition. Et donc la liaison au sein de l'article 11 de l'ordonnance statutaire de l'impartialité au droit syndical permettrait de préciser. L'étendue exacte de cette notion d'autant que la Cour européenne, droits de l'homme, je vous le rappelle protège. Très clairement, la liberté d'expression des magistrats syndiqués dans les cadres législatifs fixé. Quel est l'avis du gouvernement.

L'exercice du droit syndical des magistrats. Et la liberté d'expression qu'il implique. Doivent être concilié avec le devoir de réserve. C'est d'ailleurs ce que rappelle un arrêt récent de la Cour européenne. Ce devoir de réserve, il est prévu à l'article 10 du statut. Et il s'impose à tout magistrat. Y compris les représentants syndicaux. Je suis d'accord avec vous sur le fait que si l'exercice du droit syndical. Suppose une certaine liberté d'expression. Celle-ci bien sûr ne doit pas porter atteinte à l'image de l'autorité judiciaire afin de. Préserver la confiance. Des citoyens dans leur justice. Les modalités d'exercice de ce droit ne doivent pas davantage porter atteinte à l'exigence d'impartialité des magistrats garantie tant par la Constitution que par l'article. 6 de la Convention européenne. La frontière entre l'outrance. Parfois critiquables. Et la liberté d'expression syndicale est un sujet très sensible et qui réclame, me semble-t-il. Une réflexion approfondie. Et cette très exactement pour cette raison. Que j'ai récemment saisi pour avis. Le Conseil supérieur de la magistrature avec lequel je travaille et je veux instaurer entre le Conseil supérieur de la magistrature et la chancellerie. Des Liens qui sont déjà étroit mais qui doivent encore. Se renforcer. Donc oui, j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature de cette question de la liberté d'expression des magistrats sous les différentes formes. Qu'elles peuvent emprunter et il me semble en conséquence. Qu'il serait prématuré de toucher au statut des magistrats sur ce point avant d'avoir obtenu la réponse du Conseil supérieur de la magistrature en aucune façon, je ne veux si j'ose dire enjamber le Conseil supérieur de la magistrature, à qui j'ai demandé un avis et je sais que ce sera un avis, sage. Et un avis extrêmement important. J'ai, je suis d'autant plus prudents que nous sommes tenus au respect des normes constitutionnelles mais également. Européennes, la Cour européenne des droits de l'homme. Je viens de faire allusion à cette décision. C'est d'ailleurs positionné le 6 juin. En censurant. Une décision disciplinaire prise à l'encontre d'une magistrate. En raison de ses déclarations au nom d'un syndicat de magistrats dans la presse. Mais cet arrêt rappelle aussi le devoir de d'aisé de réserve et tout ça est un juste équilibre qu'il faut réaffirmer l'ajout vous proposez pose évidemment une question intéressante je le dis mais un peu prématurée. Je vous propose donc, Monsieur le sénateur. Un retrait dans l'attente de l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des faux je serai défavorable à votre amendement. Merci madame la présidente. Ainsi, voilà donc le retour de. L'exercice. Du droit syndical des magistrats. Et peut être même si je ne crois pas avoir vu d'amendements en ce sens, leur interdiction. Donc. Notre collègue Bonnecarrere. Souhaite indiquer respect du principe d'impartialité qui s'impose, membre du corps judiciaire. Alors évidemment, il connaît les termes de l'ordonnance du 22 décembre 58. Il sait que cette ordonnance dit que le droit syndical et garanti aux magistrats qui peuvent librement créer des organisations syndicales y adhérer exercer des mandats et pour que l'exercice de ce droit, les magistrats sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires de. Droit commun applicable aux fonctionnaires Il n'a échappé à personne peut être. Cela a-t-il échappé à certains que le garde des Sceaux a effectivement saisi il y a quelques semaines, le Conseil supérieur de la magistrature. De maintenir assez large et assez étonnante. De la conception du devoir de réserve, allant jusqu'à inclure les propos des magistrats, sur les réseaux sociaux, mais également plus étrange au cours des audiences solennelles. Alors il est certain quand on est garde des Sceaux. Ce qui ne m'est jamais arrivé. Ce qui ne m'arrivera jamais assisté à une audience solennelle ou un procureur général ou un président de de de tribunal. Dit ce qu'il pense de la politique pénale ou de la politique en matière de justice en vigueur, peut être un moment Inégalement plaisant. Mais c'est bien de cela dont il s'agit et dont vous avez saisi le CSM. Monsieur le Ministre. Alors. J'entends au fond quels qu'en soient les raisons. Je me réjouis que le ministre trouve que c'est un peu prématuré. J'espère que, d'ailleurs. Notre collègue va retirer cet amendement mais je dis attention. Parce que le retrait. Ou de, d'une manière ou d'une autre, de la liberté de l'exercice syndicale des magistrats. Beaucoup l'ont essayé beaucoup l'ont tenté, j'espère que ce n'est pas le chemin que vous voulez emprunter. Monsieur Mohamed Saïdi. Merci madame la présidente. Je voudrais vraiment sincèrement remercier notre collègue Philippe Bonnecarrère. D'avoir mis ce sujet. Aujourd'hui en discussion. Le sujet du respect du principe d'impartialité. Par. Les membres du corps judiciaire. Comme lui. Il n'est nullement question de remettre en cause. L'exercice du droit syndical ni le principe ni l'exercice du droit syndical. Des des magistrats. Et moi je, je peux comprendre les réserves. Émises par le garde des sceaux qui est dans dans son rôle. Mais lorsque. L'on regarde certaines prises d'opposition. De magistrats. Au nom. De leur syndicat. Et lorsque, par la suite. On constate les décisions prises. Par ces mêmes magistrats. J'allais dire un application. Mais de leur. Opinion. Eh bien cela a des effets dévastateurs. Parce que c'est perçu comme des prix jugement. Et lorsque l'on sait que. Les décisions de justice sont censés être rendue au nom du peuple français. Eh bien lorsque vous avez des citoyens qui ne comprennent pas, ni le sens. la, la façon dont ces, ces décisions ont été rendues. Je peux vous assurer que dans des territoires notamment les territoires reculés de de métropole, cela peut avoir des effets dévastateurs. je je demande à notre collègue de maintenir son amendement. Et je vais le voter pour asseoir ce débat quelles que soient les suites qui en résulteront. Si Monsieur le Ministre, Monsieur Bénard avant. Pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, j'aurai la parole après les explications de vote des sénateurs. Oui. Je voulais insister sur ce qu'a développé Marie-. Pierre de La Gontrie. En fait, bien entendu. Alors vous pourrez trouver toujours un certain nombre d'exemples pour aborder la thèse que vous venez de défendre Monsieur Bonnecarrere et. Monsieur. Et. Thani mais dans la réalité, on peut trouver des exemples de ce type-là, dans des tas de professions et pour des tas de fonctions. La réalité c'est ce qu'a posé. Sur la table. Madame de La Gontrie. C'est aujourd'hui ce qu'on en arrive à remettre en cause le droit. De se syndiquer des magistrats. C'est ça la vraie question. Donc il me semble que la sagesse en l'occurrence consisterait au moins à retirer l'amendement, comme l'a demandé le garde des Sceaux de telle façon à. Imaginer concevoir prévoir parce que c'est notre travail de prévoir ce n'est pas de réagir. Un phénomène qui a pu se dérouler. Il y a 15 jours il y a 3 semaines il y a un mois. Quelles seraient les conséquences aujourd'hui Monsieur Bonnecarrere de l'adoption de votre abonnement si tenté qu'il arrivait. À être poursuivi jusqu'au bout.

de Monsieur le le ministre de chez moi, j'attire l'attention je, j'ai bien compris le sens de l'amendement de notre collègue. Bonnecarrere mais là, on ouvre des brèches quand même assez béante sur. Pour neutraliser en quelque sorte de l'activité syndicale aujourd'hui les magistrats et demain qui. Donc je dis attention. Et comme cela a été rappelé là le le le le le l'activité syndicale, si je peux la résumer ainsi, est un droit fondamental dont respectons ce droit fondamental. Monsieur le garde des Sceaux, maintenant c'est vous. Madame la présidente. Il y a vraiment possible mais je l'ai dit tout à l'heure. C'est un sujet difficile. Aucun sujet n'est tabou. Il faut regarder les choses avec calme et et auteur. J'entends bien. Madame de La Gontrie, que vous ne serez jamais garde des Sceaux, méfiez-vous. J'ai dit ça aussi Oui oui mais je je je sais mais. Vous, peut-être que vous le voulez, je n'en sais rien mais mais, méfiez-vous. Méfiez-vous de ces postures. On est parfois pris ensuite. À ce qui semble être un piège. Je je veux rappeler les choses. Je vais le faire vite. Voilà le recueil des obligations déontologiques des magistrats. On peut y lire que le magistrat. Dans son expression publique doit faire preuve de mesure afin de ne pas compromettre. L'image d'impartialité. De la justice, indispensables à la confiance du public, ce sont les mots que j'ai repris tout à l'heure. Dans ma réponse. Cette exigence rajoute. Le premièrement du chapitre 8 s'impose, quel que soit le moyen de communication. Même madame la sénatrice. Les réseaux sociaux naturellement. Deuxièmement et puis je m'arrête là, ensuite. Et chacun appréciera. Toute manifestation d'hostilité aux principes et à la forme du gouvernement de la République est interdite aux magistrats. De même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction. Maintenant. Vous avez évoqué cette lettre, je vais vous en communiquer la teneur. Parce que ça me paraît important. J'ai adressé effectivement le le 2 mai 2023. Au Conseil supérieur de la magistrature. Un courrier. Dans le 1er, grave, je, je rappelle que nous sommes. En train de travailler sur. La suite des états généraux. Je je je le passe j'évoque dans le 2ème paragraphe un 3ème grade. On l'évoquera, bien sûr, la rénovation des modes d'accès à la magistrature. Et puis j'en viens au fait qui nous intéresse à cet instant. J'écris en pleine concertation avec le Conseil. Je souhaite continuer à approfondir la réflexion sur le statut de la magistrature. Avec l'objectif de toujours mieux préserver l'image de la justice aux yeux de nos concitoyens. C'est pourquoi je sollicite l'avis du Conseil sur les 2 points suivants. Ces dernières années. Les réseaux sociaux sont devenus un vecteur important si ce n'est le vecteur principal d'information de nos concitoyens. Les chefs de juridiction et de cours et notamment les procureurs de la République ont massivement investi ces plateformes afin de toucher les Français et de leur faire découvrir le quotidien des juridictions ou communiquer sur les affaires en cours. De plus, de nombreux magistrats ont créé des comptes sur divers réseaux sociaux anonymes ou non et s'en servent pour commenter l'actualité judiciaire, juridique et politique. Ou plus prosaïquement pour partager des événements de leur vie privée. Cet usage des réseaux sociaux et l'importance croissante qu'ils ont pris dans le débat démocratique bouscule le traditionnel équilibre entre la liberté d'expression reconnue à chaque magistrat et l'obligation déontologique de réserve et de discrétion. De manière plus générale les formes de plus en plus diverse que revêt l'expression publique individuelle ou collective de magistrats à l'occasion d'audience solennelle ou encore par le biais de l'expression syndicale peuvent parfois pour pour l'opinion publique. Interrogé, le respect des obligations de réserve et de neutralité, ainsi que des règles déontologiques et donc nuire à l'image de la justice de manière générale la conciliation entre les libertés individuelles et collectives des magistrats et le respect de leurs obligations déontologiques m'amène également à solliciter votre avis sur la conformité avec le statut de l'exercice du droit de grève, c'est un autre sujet mais je tenais à préciser les mots qui ont été utilisés pour saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Je suis gourmand d'avoir son avis et il, mais je le dis indispensable. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté un amendement 74 présenté par le gouvernement. Merci madame la présidente. C'est c'est très simple à résumer cet amendement s'agit de créer un accès à la magistrature dédié au Docteur en droit.

Dans le même esprit que l'article 78 de la loi à 2013 660 du 22 juillet 2013. Qui contient plusieurs mesures consacrés à l'insertion professionnelle des docteurs notamment à l'amélioration de l'accès des docteurs, la fonction publique. La rédaction actuelle se référant au grade nous paraît être source de confusion entre le diplôme du doctorat à lui-même le titre partagé par les titulaire de plusieurs diplômes et le grade susceptibles également d'être partagé par les titulaire de plusieurs diplômes de statuts différents. C'est cette confusion que nous présentant qui risque d'aboutir à une moindre valorisation du diplôme. Ce qui pourrait être le résultat inverse de celui qui est recherché par le l'amendement que nous soutenons du gouvernement. Le comité des états généraux de la justice 2022 piloté par Jean-Marc Sauvé regretter l'absence de dispositif de recrutement adapté à la recherche de profils de haut niveau comme la lenteur et la cohérence du processus de recrutement latéral. Or ce type de recrutement pour être un moyen de favoriser l'intégration de profils très spécialisés dotées de solides connaissances dans certaines branches du du droit pour compenser. Les déficits relevés en juridiction la rédaction proposée dans le sous-amendement explicite à la fois que ce sont bien les titulaires du diplôme national du doctorat qu'il s'agit de valoriser pour l'accès à la magistrature et à la fois de prévoir un parcours adapté à leur niveau de formation au lieu d'en les dispensant des épreuves d'admissibilité. Je vous remercie. Elle est l'avis de la commission sur cet amendement et ce sous-amendement. Ont été un peu oubliée dans la modernisation des voies d'accès prévu à l'article 1 du projet de loi organique. On avait eu ce débat en commission, nous avions cherché des solutions le gouvernement en propose une, qui, qui est d'ailleurs complémentaire de celle que nous proposerons, par la suite parce que dorénavant, il y a deux formes d'accès pour essayer de simplifier cette question des voies de recrutement. Une forme d'accès via l'auditorat donc avec une formation de 31 mois à la clé qui concernent soit des recrutements donc d'étudiants de voies interne ou externe ou interne ou une voix du du 3ème concours c'est ce troisième concours que souhaite étendre le gouvernement au. Doctorant qui ont un autre diplôme d'études supérieures et nous y sommes favorables par contre Monsieur Ben arrange tout amende en voulant dispensés d'épreuves d'admissibilité pour les deux les docteurs on ne voit pas pourquoi on. Dans cet objectif de simplification, on trouverait une X ième voix différentes, pour les docteurs concours. Ministre quel est votre avis sur le sous-amendement de monsieur Bena Roche. Je préfère mon amendement madame la présidente. Je suis des je suis défavorable au sous-amendement de monsieur. Très bien je vais donc mettre aux voix d'abord le sous-amendement de monsieur Bena Roche qui est pour qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je mets maintenant aux voix l'amendement du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Nous passons maintenant à 2 amendements identiques. Je ne commence par le 7. Madame de La Gontrie. Merci madame la présidente. Il s'agit simplement de garantir que. Les places offertes au titre du concours étudiant le 1er concours. Soit au moins de 50%. Merci. Le 47, madame Assassi. Oui merci madame la présidente. Il s'agit exactement du même abondement que précédemment défendu. Quel est l'avis de la commission. Ce sera un avis défavorable. En effet, vous voulez que le nombre d'auditeurs recruter au titre du 2ème concours et du 3ème concours ne peuvent dépasser la moitié ne peuvent au titre des 3 concours pour l'auditorat. Donc le but c'est effectivement. De augmenter le concours étudiant qui doit oeuvrer représenter selon vous au moins la moitié des places, nous ne sommes pas favorables, en fait, on pense que les craintes que sous-tend votre amendement sont disproportionnées. On a fait le, le ratio d'un tiers pour le recrutement au titre du 3ème concours est issu de l'ancien ratio désintégration sur titre. Il se justifie par la suppression de certes de cette voie d'accès dont les candidats devraient naturellement se déverser vers le concours. Professionnel, vie des candidats n'ayant pas vocation à connaître une évolution massive des ratios de recrutement entre les étudiants, fonctionnaires et professionnelle devrait en réalité être identique en second lieu, il convient à notre avis de ne pas rigidifier et les structures de recrutement. Nous sommes plus favorable à une grande ouverture. Du corps judiciaire sur le monde professionnel. C'est pourquoi nous émettons un avis défavorable. Ah ces deux à Monsieur le Ministre même même avis. Je mets Je mets aux voix ces deux amendements identiques double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Ils ne sont pas adopté 3 amendements en discussion commune. On commence par madame présenté pour le 53 à monsieur Ouzoulias pardon. Merci madame la présidente, monsieur le le garde des Sceaux je je reviens sur ce problème du du doctorat en droit. Il y avait une une passerelle depuis 1958 qui permettait au Docteur en droit et uniquement à cela de devenir des auditeurs de justice et pour ce qu'il avait 3 ans d'expérience professionnelle de de pouvoir devenir juriste assistants. C'était une voix très importante parce qu'elle donnait de la valeur au doctorat en droit et elle permettait d'accéder à, à ces professions. Vous supprimez cette passerelle ce dispositif. J'ai bien entendu Monsieur le Ministre, que vous ouvriez une une 3ème voie mais ça n'a pas tout à fait la même valeur, et ce que je crains c'est que avec ce dispositif il y a une forme de dévalorisation de du doctorat en droit. Or. Dans ce même hémicycle. Lors de la loi de programmation de la recherche. Nous avions tous dit de façon unanime que la France se caractériser dans le contexte européen par une faible attractivité de son doctorat et notamment par le fait que il y a peu. Docteur dans l'administration et dans les services publics. Contrairement à l'Allemagne à l'Allemagne où ils sont beaucoup plus présents. Ce que, ce que je crains avec avec cette suppression c'est que malheureusement il y a une perte d'attractivité de du doctorat en droit. les professeurs. Nous disent et c'est un peu contradictoire par rapport à la politique que vous menez. Par ailleurs, de revalorisation. Du diplôme de Docteur, merci madame la présidente. Monsieur Bena arrange pour l'identique il est défendu. Très bien défendu par monsieur Julia. justement pour pour permettre. De réintroduire c'est, c'est pas exactement le même pour obliger de réintroduire la procédure 18. Permettant au Docteur en droit. D'accéder à une formation longue de 31 mois par le biais d'une nomination directe en qualité d'auditeur de justice. C'est ce qu'a dit très bien monsieur Julia. Parce qu'en fait nous ce qui nous perturbe en en fait en dehors de ça, c'est que le les les deux voies qui sont ouvertes actuellement c'est le concours professionnel mais c'est avec une formation courte. Ou le 3ème concours qui est limité par un quota. promotions. La richesse des promotions expliqué par mon collègue Ouzoulias. Réduite sur la voie d'accès au 18, à part le nouveau dispositif ne permet pas en plus pour ceux qui le souhaiteraient, d'avoir accès à une formation longue. C'est ça aussi que nous déplorons. Il y a les deux, il y a le fait qu'on puisse plus à avoir accès à cette richesse de 18 et en plus qu'on ne puisse puisse choisir une formation longue puisque la seule ouverte. Ce serait une formation courte. Merci. Quelle est la ville la commission sur ces deux amendements de 53 et 36 le n'ayant pas été défendu. Alors effectivement ils sont pas totalement identiques mais quand même très proche. Ce sera un, un, un, un avis pardon défavorable. En effet ces deux amendements tendent à restaurer la voie d'intégration directe à l'ancien second grade, notamment pour permettre aux docteurs d'en bénéficier. Nous sommes plutôt favorables à l'unification des voies d'accès, telle qu'elle est proposée aujourd'hui et donc qui ne permet plus cette intégration directe mais qui ouvre d'autres voies dont on vient de parler et d'autant plus que nous

donc défavorable à la réintégration directe. Monsieur le garde des Sceaux même avis. C'est même position défavorable. Madame la présidente. Je mais aux voient d'abord l'amendement 53 double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté le 36 même vote.

Madame Canayer. Donc je pense que je vais faire assez court. C'est la possibilité d'intégrer les docteurs en droit à la voie d'accès au concours professionnel pour combler une partie du manque. Que nous n'avons pas réussi à combler dans l'amendement précédent. Voilà mais je laisse Madame Canayer développer.

pour les docteurs. Cela à la suite aussi de la réforme de l'INS P. C. T. l'intention initiale du gouvernement et on pense que la proposition du gouvernement et la nôtre est identique à celle de Monsieur Bénard roches sont complémentaires. Quel est l'avis du gouvernement sur ces deux amendements. Même avis madame la présidente. Donc vous avez avis favorable c'est difficile de se caler sur son avis. Donc pour vous, Daniel votre vous avez raison, je les expliciter pardon. Le concours professionnel il se destine aux professionnels qui justifie d'une expérience particulièrement qualifiantes. Pour être magistrat puisque la formation qui leur sera dispensée sera plus courte. Et c'est la raison pour laquelle les durées d'activité professionnelle qui sont demandées aux candidats pour se présenter. Sont réduites pour les professionnels ayant une activité très proche de la sphère judiciaire. Je pense aux avocats ou juristes assistants s'attacher justice au directeur de service de grève. Telle n'est pas le cas des docteurs en droit. Quand bien même quand bien même il justifierait de 5 années d'enseignement ou de recherche. Situation des docteurs en droit. Cependant pas été omise d'autres voies d'accès leur sont offertes. Leur permettant de bénéficier d'une formation. Plus longue. Les conditions vous proposez pour leur ouvrir la voie du concours professionnel leur permettent d'ores et déjà de présenter le 3ème concours je vous propose d'ailleurs, pour tenir compte de la spécificité du parcours des docteurs en droit. Un amendement qui vise à rétablir une voie d'accès spécifique à ce 3ème concours pour les docteurs en droit. Titulaire d'un autre diplôme d'études supérieures et qui ne justifierait d'aucune expérience professionnelle et pour l'ensemble de ces raisons je suis défavorable à cet amendement. Voilà. Je vais donc mettre aux voix, ces deux amendements identiques, dont un de la commission qui ont reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Ils sont adoptés. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 33 de madame de La Gontrie. Merci madame la présidente. à ce stade du projet de loi organique vous proposer un dispositif intéressant qui permet et c'est un petit peu votre quête à travers l'ensemble de ce texte. De recruter des magistrats de meilleur niveau possible évidemment. Et de ce fait d'ouvrir le plus possible les accès. Latéraux. Sauf que. Il nous a semblé que ce qui était permis par exemple aux avocats. Le calendrier qui était prévu en terme de formation et de probation n'était pas compatible avec la réalité de l'exercice d'avocats. Je m'explique. Si j'ai bien compris le dispositif que vous que vous développez dans cet article, Monsieur le Ministre. Il y a. Un une première sélection en quelque sorte, puis un stage probatoire et à l'issue duquel vous pouvez ne pas être retenue. Mais ce stage probatoire dure 12 mois. Donc je ne sais pas comment, lorsqu'on est avocat, on peut mettre en sommeil son activité pendant 12 mois, sachant qu'à l'issue, on peut ne pas être. C'est pour ça que nous proposons un mécanisme en 2 temps. Un stage probatoire effectivement qui permettrait de ne pas retenir le candidat mais limité à 3 mois et quand même une formation ensuite. Jusqu'à l'obtention de de l'intégration qui elle nous proposons qu'elle soit portée à 15 mois en tout donc il ne s'agit pas d'en d'en rabattre sur la qualité des personnes recrutées mais si nous voulons. Je pense que c'est votre objectif que cette filière soit attractive il faut que cela puisse correspondre à à la réalité et je rappelle que 3 mois, ce sont des durées qu'on pourrait qualifier de manière un peu rapide de période d'essai, mais c'est une durée qui permet, me semble-t-il d'évaluer si la personne postulante est absolument inadaptés à la fonction qu'elle envisagent d'occuper.

Merci madame la présidente. Avoir les moyens d'embaucher, c'est une chose, pouvoir le faire évidemment s'en est une autre. Alors d'abord saluer le le le travail qui a été réalisé par. Mesdames les rapporteurs et dont j'ai adopté. Évidemment, un certain nombre de propositions. Mais je ne peux que m'opposer certaines évolutions proposées par la commission des lois. Certains des rétablissements qui nous sont demandés sont d'ordre exclusivement. Juridique. D'une part fixer la composition des jurys relève du pouvoir réglementaire. Aucun des différents jurys qui existe actuellement n'est défini dans la loi organique. Vous souhaitez prévoir que le jury soit minoritairement composée de magistrats. Or ce jury est un jury d'aptitude et non un jury de recrutement. La présence de magistrats en nombre suffisant. Paris donc nécessaire. Et je rappelle que le jury d'aptitude est aujourd'hui composée en minorité de magistrats aujourd'hui 4 sur 9. Il y a donc aucune raison que ça change. Je souhaite donc en conséquence que le Champ du pouvoir réglementaire soit respectée. Pour ne pas instaurer ce type de limite. Quant à la proposition de magistrat détaché, il y a un risque de censure constitutionnelle. Qui ne justifie pas d'être pris puisque nous sommes très loin d'atteindre le quota actuellement autorisés et validé par le Conseil constitutionnel, La précision apportée quant à l'interdiction pour les magistrats en service extraordinaire. D'être nommé membre du jury d'aptitude des stagiaires est inutile, juridiquement il n'entre pas dans la définition que fait le Conseil constitutionnel de l'expression magistrats de l'ordre judiciaire. C'est surtout la question de la durée de la formation des stagiaires. Que vous souhaitez encadrer au niveau organique qui me pose, je le dis, une vraie difficulté. Alors qu'un tel niveau de normes n'est pas requis. Aucune durée de formation n'est précisé dans la loi organique, qu'il s'agisse des auditeurs de justice des candidats à l'intégration ou des lauréats des concours complémentaires. Je ne vois aucune raison de de déroger à cette règle et ce d'autant moins que le gouvernement a indiqué en toute transparence, qu'il envisageait une durée qui ne serait pas inférieure à 12 mois pour l'exercice de fonctions. Généraliste seulement. Une durée de formation de 18 mois ne permettra pas au gouvernement de tenir son engagement et je le dis de recruter 1500 magistrats dans le délai qu'il s'est fixé. Alors c'est quand même le but de ce texte, je l'ai dit les moyens oui ensuite si on permet pas de recruter les magistrats. On n'a pas apporté ce souffle dont notre justice a tellement besoin et c'est la raison. Essentielle pour laquelle je vous demande de faire droit à cet amendement de rétablir certaines dispositions du projet du gouvernement, sinon nous aurons du mal à tenir. Nos engagements et nos engagements. Je je je peux vous dire pour être toutes les semaines en juridiction qu'ils sont particulièrement attendues dans leur réalisation concrète d'ailleurs pour ne rien vous cacher. Souvent j'entends des greffiers des greffières des magistrats qui me dit mais qu'est-ce qu'on fait en attendant que le texte. Soit voté qu'il soit applicable et vous savez ce que je réponds, je réponds, il faut patienter patienter encore un peu. C'est dire les attentes que suscite ce texte il faut que. Nous puissions mettre en application et en Oeuvres ce que tous ensemble nous voulons faire. Madame la rame. L'amendement huit étant défendu madame la rapporteure. Quel est votre avis sur ces trois amendements.

Merci à la présidente. Alors sur cette discussion commune sur les trois amendements concernant la durée enfin et l'organisation du, du recrutement et de la formation des stagiaires. Donc ce qui. Relève du concours professionnel. Alors pour l'amendement 33 de Madame, Aribi, Aribi, cet amendement prévoit que la formation des stagiaires serait porté à 15 mois. Cela reviendrait à diminuer la durée de formation proposée en commission puisqu'en commission, je vous rappelle que nous avons, au moins 18 mois, avec notamment une augmentation et c'est pour répondre à monsieur le garde des Sceaux. De la période du stage d'application en juridiction et donc ces stagiaires parce que effectivement on comprend l'enjeu de recruter 1500 magistrats ont c'est comme vous, comme ils sont attendus dans les juridictions, ça fait plusieurs années qu'on a ces débats au moment de la loi de finances 2, néanmoins suffit aussi enfin il est important aussi que les magistrats soient bien formés et que une fois qu'ils arrivent en juridiction il soit il faisait. et les compétences suffisantes. C'est pour ça. Que nous proposons une formation d'au moins 18 mois avec une extension du stage de pré-affectation en juridiction. Alors c'est vrai que il y a. Un sujet qui nous ont été relevés pendant les auditions. Elle ont insisté Madame arriver et madame de La Gontrie. C'est la situation des avocats notamment ou de chefs d'entreprises qui passe le concours et qui doivent laisser leur activité professionnelle pendant la durée. De leur formation et qui ont toujours un risque, si jamais ils ne sont pas acceptés par le jury. Eh bien ils risquent de perdre leur activité professionnelle donc ça allait mais dans une forte C'est pourquoi nous vous proposerons par la suite un amendement qui vise à adapter effectivement les conditions de la formation à la situation professionnelle. Des stagiaires

Supprimée enfin ou modifier largement pardon plutôt en commission je reviens pas sur la durée de la formation, je viens de vous en expliquer les les raisons sur la composition du jury. Nous pensons que même si ça résiste de du niveau réglementaire que nous avons quand même la capacité de fixer un cadre. Dans la loi organique, c'est pour ça que pour éviter tout risque de corporatisme, nous prévoyons que les jurys ne peuvent comporter une majorité de magistrats et cette. Le rôle et enfin sous s'agissant de l'ouverture de la proportion de magistrat détaché certes le quota d'un vingtième n'est pas. Atteint mais c'est pas une raison pour ne pas l'ouvrir parce qu'on pense que c'est une bonne chose d'avoir des magistrats détachés. Et donc nous sommes favorables à un quota de 1 quinzième. Donc. Voilà. Et pour la la donc un avis défavorable sur l'amendement du gouvernement et enfin sur l'amendement numéro 8 de Madame Harribey. Nous pensons que. Pareil, ça remet en cause ce qui nous a adopté sur la composition du jury professionnel. Donc nous sommes aussi défavorable. Je suis défavorable aux deux amendements le le 33 et le et le numéro 8. Je voudrais dire. Qu'aujourd'hui pardon. Défavorable.

si je peux si je puis me permettre hein le rapporteur. Vous m'avez pas répondu sur le volet formation. Le temps de formation c'est c'est ce qui inquiète. Non mais je je je le dis, c'est ce qui inquiète beaucoup ceux qui aujourd'hui envisagent d'entrer dans la magistrature. C'est un énorme sujet d'inquiétude. Et si le durée de la, la durée de formation parce que vous parlez d'excellence oui bien sûr. Je rappelle qu'il y a un jury qui aura une évaluation que. Ceux qui ont exercé le le le métier d'avocat à la profession d'avocat pendant de nombreuses années sont aptes. Évidemment et et. Je je je le redis, c'est pour nous une question cruciale, il faut permettre. D'élargir ses passerelles qui sont aujourd'hui beaucoup trop étroite à mon sens. Bien je vais donc mettre aux voix. Monsieur Richard, monsieur le président Richard. permettent de d'apporter mon soutien au garde des Sceaux mais mais un. Un soutien seulement partiel. Je crois qu'il est. Tout à fait soutenable endroit. Que l'idée. D'une majorité non magistrats dans le jury relève bien du niveau organique puisque ça. Consiste vraiment à encadrer les conditions d'accès à la profession. Malheureusement je pense que sur le fond, cet amendement. Inopportun. Car comme l'a dit le garde de façon tout à fait clair, il s'agit cette fois-ci d'apprécier directement la capacité à exercer en juridiction et donc la présence en quelque sorte moral de personnes qui ne sont pas des professionnels de l'activité juridictionnelle et ne peut être que minoritaire en revanche. Je crains monsieur le Ministre, parce que c'est une. C'est une habitude. Assez fréquente quand même. Dans le monde parlementaire de vouloir transgresser de traverser la limite entre le législatif et réglementaire mais je me permets de rappeler. Au gouvernement qui n'en fait pas usage qui lui une procédure de déclassement.

au moins 18 mois, on ne touche pas à la partie théorique simplement n'allonge le stage de pré-affectation pour qu'il se forme plus auprès de leurs confrères dès, dès lors qu'ils sont déjà affectés dans leur juridiction, donc ça permet quand même. De remplir leur fonction. Ça permet quand même de. De de permettent. De de viser les recrutements dont vous avez besoin et ça permet aussi de garantir une qualité de la formation pour ces magistrats stagiaire.

Même vote. Il n'est pas adopté et madame la rapporteure. Vous avez la parole pour 78. en fait le régime des stages et d'études en fonction de, le, la formation d'origine de l'expérience professionnelle ou le cas échéant de la poursuite de l'activité professionnelle des stagiaires. Istres, qu'en pensez-vous. Merci madame la présidente, madame. La rapporteure. L'joue vous proposez qui concerne la possibilité pour un stagiaire issus du concours professionnel. Me paraît incompatible. Avec leur statut. Je ne peux pas être plus clair en 1er lieu parce que. Cette formation dont la durée envisagée par le gouvernement fait l'objet de critiques ne peut pas être envisagé comme une formation. Qui ne serait pas à temps plein et donc adaptée pour permettre un cumul d'activité et cette règle vaut d'ailleurs pour tous les fonctionnaires stagiaires qui doivent se consacrer entièrement à leur formation et il en va de même pour les magistrats. Tous les stagiaires seront rémunérés pendant l'intégralité de cette formation et de plus. J'imagine difficilement qu'un avocat puisse effectuer son stage juridictionnel en même temps qu'il poursuit son activité libérale. Même en dehors du ressort et sans faire naître un risque de conflit d'intérêts et je rappelle enfin que le statut de la magistrature prévoit divers statuts qui permettent l'exercice à temps incomplet des fonctions de magistrats et qu'en pareille hypothèse un cumul avec une autre activité professionnelle est possible. C'est notamment le cas des magistrats à titre temporaire qui bénéficie qui bénéficie en outre d'ailleurs d'une voie d'intégration définitive dédié l'intégration de la magistrature doit être un véritable choix. En conséquence je suis mais. Viscéralement opposé à cet amendement. Une fois n'est pas coutume je partage absolument le l'avis du garde des Sceaux. On est dans une prise de risque maximale. C'est d'ailleurs pour ça qu'il eut fallu voter mon amendement 33. non mais c'est intéressant de voir comment vous tournez autour du problème, comment faire pour qu'un avocat qui exerce puisse changer de voie professionnelle sans pour autant mettre en péril son activité si par hasard ça ne se Nous avions proposé une voix vous ne l'avez pas voulu en estimant que la vôtre était meilleur sauf que là la votre n'est pas acceptable. Donc. De ce point de vue, je pense qu'il y a une vraie prise de risque et je pense que vous devriez le retirer. Et si nous faisions plus court et à temps plein. Plus court et à temps plein. Malheureusement je ne peux pas remettre au vote l'amendement précédent madame de La Gontrie. Et donc je vais donner la parole à Madame la rapporteure.

pendant une période de formation trop longue qui met en péril leur activité professionnelle. On pense que. La solution proposée par Madame de contre ils n'étaient pas satisfaisantes parce qu'elle crée aussi des systèmes qui était trop dérogatoire Nous on a une solution qui est plus large, peut être. Qui permet d'adapter, elle est certainement pas satisfaisante. Peut-être que nous devons profiter de la navette pour pouvoir trouver une solution efficace en la matière. Très bien. Très bien. Nous passons maintenant à l'amendement numéro 9 de madame de La Gontrie. Gérard Clément.

Même avis jamais aux voix double avis défavorable. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 56. Il n'est pas défendu, je me vois l'article 1er qui est pour. Qui est contre qui. Explications. je vous donne la parole pour une explication de vote santé 1er. Je souhaitais faire une explication. De vote rapide. Je n'ai pas voulu revenir tout à l'heure sur. Les échanges avec le garde des Sceaux avec plusieurs d'entre vous sur la question de l'impartialité. Je réexprime en quelques secondes votre point de vue. Nous pensons que la question de l'impartialité est au coeur de la vie de la démarche et de l'action des magistrats que cela soit dans leur action individuelle ou collective. Nous sommes conscients des enjeux de l'action syndicale et la liberté d'expression au monde, donc de manière classique. À trouver un équilibre entre pour reprendre les formulations habituelles du Conseil constitutionnel entre 2 objectifs à valeur constitutionnelle, monsieur le garde des Sceaux le et vous avez eu la courtoisie de me communiquer une copie de votre courrier. La démarche que vous avez entreprise auprès du CSM pour être mieux informés pour reprendre votre formule Dominique judiciaire sa sagesse sur ces questions, nous espérons très simplement que d'ici la fin de la navette, nous ayons la réponse du CSM et nous entendions et nous Nous avons maintenu notre amendement pour que la discussion puisse avoir lieu que ceux-ci restent dans le débat mais nous partageons votre souci d'équilibre Comment dire le, l'approche commune d'une particulière sagesse dès que l'on touche au monde de la justice. Merci. S'il n'y a pas d'autres explications de vote sur cet article premier, je vais le mettre aux voix qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. Nous passe ensuite l'amendement 34 n'est pas défendu, nous passons donc aux 52 de madame la présidente à. merci madame la présidente. En fait, avec cet amendement, nous voulons insister sur la nécessité de garantir une représentation majoritaire des magistrats au sein du collège d'évaluation et c'est pourquoi nous proposons que les magistrats occupe une position majoritaire au sein du collège, tout en permettant la présence de personnalités qualifiées ayant une expertise spécifique en matière de gestion des ressources humaines ou ou budgétaire et donc c'est à moi, cet amendement prévoit que ces personnalités qualifiées ne représente pas plus de 25% de l'effectif total du collège. Nous considérons en effet que l'inclusion de personnalités qualifiées apportant des conseils des compétences spécifiques complémentaires est pertinente car cela peut contribuer à éclairer les décisions du collège dans des domaines particuliers. Cependant, il nous pensons aussi qu'il est essentiel de préserver la prépondérance des magistrats au sein du collège car bien évidemment, il posait posait elles et eux l'expertise juridique et l'expérience nécessaires pour évaluer les performances et les compétences. Des magistrats. Madame de La Gontrie. Défendu. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements. Alors nous abordons ici l'évaluation à 360 degrés des chefs de juridiction et des chefs de cour. Nous considérons que

nous sommes favorables à ce que nous avons adopté évidemment défavorable aux amendements. car la commission a précisé que le collège d'évaluation doit être composé pour 25 à 50% de personnalités extérieures. Dans l'évaluation à 300. 30 degrés il y a non seulement il y a l'évaluation des capacités à gérer des capacités administratives des magistrats mais aussi leur capacité à gérer les relations avec je dire l'hinterland du magistrat du chef de juridiction et notamment dans ses rapports avec les autres. Personnalités les autres institutions. D'ailleurs j'en profite pour dire que Madame Gatel avait déposé un amendement qui n'a pas été soutenue mais que nous je suis défavorable d'ouvrir dans la formation des magistrats un stage en collectivité territoriale. Nous pensons au contraire que ce lien avec les collectivités territoriales auxquelles nous sommes attachés aussi ici au Sénat, doit être intégrée par les chefs de juridiction et que de cours pardon et que cela sera un des éléments, notamment de l'évaluation à 360 degrés et donc pour nous, il est nécessaire d'ouvrir ce collège sur l'extérieur. les chefs de cour et chefs de juridiction pour résumer doivent être davantage en prise avec la société civile. Oui, ce que vous dites madame la rapporteure est d'autant plus vrai en réalité. Que. Les juridictions les chefs de de cour et de juridiction nous demandent davantage. De déconcentration et donc il y a des choses que vont faire les chefs de cour et les chefs de juridiction qu'il ne faisait pas autrefois et il est de l'intérêt de tous et d'abord de l'intérêt du justiciable que ces choses soient bien faites. J'indique d'ailleurs que cela est cohérent avec. Un décret que j'ai signé il y a quelques jours, qui autorise désormais à ce qu'un quart du corps enseignant à l'ENM ne soit pas magistrat. peut être mais vous voyez. On peut envisager que des élus. Viennent expliquer ce que c'est que la fonction d'élu. On peut tout envisager que des chefs d'entreprise. Viennent parler de leur réalité économique. Bon l'École nationale de la magistrature est une école absolument merveilleuses, mais oui on a intérêt à ce que les choses. tu davantage ouverte vers l'extérieur mais de la même façon, j'ai demandé aux auditeurs qu'ils aillent dans les points justice à la rencontre de nos compatriotes les plus défavorisés, les plus démunis ça possède aussi de la même volonté d'ouverture et ce que je souhaite rajouter avant de naturellement vous dire que je suis défavorable aux amendements, c'est que dans l'évaluation des chefs de cour qui n'existait pas. Nous avons d'abord préparer ça avec le Conseil supérieur de la magistrature et quand je disais tout à l'heure que je souhaitais que le Conseil supérieur de la magistrature travaille davantage avec le ministère ou que le ministère travaille davantage avec le Conseil supérieur de la magistrature, c'est une réalité parce qu'effectivement, c'est comme ça que nous avons envisagé à titre expérimental dans un premier temps la notation des chefs de cour qui n'était pas évaluer. Voilà et je pense que ces choses vont dans le bon sens et dans le sens d'une d'une ouverture. Oui absolument et qui me paraît aujourd'hui absolument nécessaire est absolument indispensable. Bien je vais donc mettre aux voix, ces deux amendements qui ont reçu un, un double avis défavorable, le 52 qui est pour. Qui est contre qui s'abstiennent n'est pas adopté et j'imagine même vote sur le 10. Et nous passons à l'amendement 11 de madame de La Gontrie. Il est défendu donc qu'en pense Madame la rapporteure. Défavorable. Monsieur le Ministre même ma vie ma vie qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Monsieur Cabanel, c'est vous qui prenez-le. Le trois, il est défendu. Quel est l'avis de la rapporteure favorable, Monsieur le Ministre même avis. Même vote n'est pas adopté et le 79 qui est un amendement rédactionnel de la rapporteure si Monsieur le Ministre, n'y voit pas d'inconvénient et l'Assemblée non plus, on peut considérer qu'il est également adopté il y a-t-il des explications de vote sur l'article 2. Je n'en vois pas, je le mets donc aux voix qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté. Nous passons maintenant à l'article 3 avec l'amendement de. Monsieur Cabanel il est défendu. Très bien. Le 14. Madame de La Gontrie. Il est défendu aussi bien qu'elle ait l'avis de la commission sur ces deux amendements défendus avis défendu. Défavorable dans les 2 cas Ministre même avis. Je ne sais pas, je ne veux pas présumer. D'accord je mets donc on voit ces deux amendements le de double avis défavorable pour qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté. J'imagine le même vote sur le 14 Et nous passons à deux autres amendements dont Monsieur le Ministre, l'amendement sont 9 du gouvernement qui n'est pas défendu, vous allez défendre. Le président de la commission mesdames les rapporteurs mesdames et messieurs. Sénateur cet amendement il tend à supprimer les durées minimales. D'exercice des fonctions. La durée maximale d'affectation dans la même juridiction. Qui ne sont pas justifiées. La magistrature est un corps particulièrement mobiles. Et nous cherchons à en limiter les effets par des lignes directrices de gestion. Le système qui est actuellement en place repose sur un dialogue nourri. Entre la direction des services judiciaires. Et le Conseil supérieur de la magistrature et ça fonctionne. La solution que vous proposez, source de rigidités. Que les dérogations envisagées ne permettent pas de couvrir. Qu'est ce que l'on fait par exemple. D'un magistrat. Qui après un peu plus de 2 années d'exercice serait candidat retenu un détachement. Je dois dire non. Alors qu'il est. Possible. Qu'il aille qui possède les compétences particulières en adéquation avec ce poste. Et ce au seul motif qu'il n'a pas exercé 3 années dans ses fonctions. Pardon de dire que ça n'a ça n'a pas de sens.

Oui peut-être mais ils sont encore plus utile auprès du garde des sceaux qui le conseille. Tous les jours. Que dire. J'ai une autre question simple pragmatique pratique. Que dire à un magistrat qui faisant face à des difficultés médicales. Souhaite se rapprocher de son lieu de prise en charge mais il a pas fait ces 3 années d'affectation et ce qu'on lui dit. On le dit, tant pis. Donc il faut que les choses soient un peu plus souple. La gestion des ressources humaines des magistrats à l'instar de ce qui est prévu dans les autres corps de la haute fonction publique nécessite de mon point de vue une appréhension des situations individuelles au cas par cas. Et sur la base de lignes directrices de gestion. Il y a pas lieu de traiter différemment les mains les magistrats des autres corps. Et ce d'autant plus que les magistrats sont. Au terme de l'article 64 de la Constitution inamovible et que les entorse à ce principe, ont toujours été motivés et validé par la volonté de préserver l'impartialité des magistrats. Si c'est l'effet d'aubaine dans l'accès au 3e grade que vous cherchez à supprimer, alors que les évolutions. Que ce projet de loi propose quant à la structure du corps. Judiciaire. Cela tente. Tendant à limiter en offrant d'autres perspectives. Je suis enclin à proposer une évolution permettant de faire disparaître et moins attentatoire au principe d'inamovibilité. Enfin ériger la règle de 10 ans d'affectation minimale me semble contraire au principe constitutionnel d'inamovibilité la limitation actuelle sur les fonctions spécialisées imposent aucunement une mobilité géographique mais simplement un changement de fonction, y compris au sein du même Je demande en conséquence de faire droit à cet amendement. Il est défendu. Donc madame la rapporteure a donner son avis sur ces deux amendements. Je vais le défendre alors. Pour ce qui concerne l'amendement 69 du gouvernement. Si nous avons souhaité mettre des conditions minimales et maximales d'affectation dans les juridictions, c'est bien parce que nous avions aussi des raisons premières remarque monsieur le garde des Sceaux. On ne peut pas légiférer sur la base d'exception et sur la base de cas qui sont à la marge, une règle de droit, on a toujours appris qu'une bonne règle de droit, c'est une règle qui a des exceptions et que dans la loi, on doit mettre le principe et qui vous a permis drap après par la voie réglementaire, vous nous l'avez dit tout à l'heure d'en définir les modalités et les limites. C'est une première chose. Si nous avons mis ces bornes de 3 ans et de 10 ans. Trois ans minimum d'affectation 10 ans maximum d'affectation. C'est pas parce que c'est sorti du chapeau et que ça nous a paru l'idée du siècle mais c'est bien parce que ça correspond à un besoin. La durée minimale, ça correspond aussi. À ce qui nous ait a été présentée à de nombreuses reprises dans des auditions. Par l'ensemble des acteurs, éviter les risques d'aubaine notamment par l'accession au 3e grade pour les chefs de juridiction. Qui. A prendrait cette fonction de chef de juridiction et se mettrait illico Presto en détachement. Une fois qu'ils auraient acquis ce 3ème grade donc l'affectation de trois ans minimum répond à cet objectif, l'affectation de 10 ans maximum. Elle vise à garantir l'impartialité des magistrats et éviter aussi tout en respectant, dans un souci d'équilibre. Ce principe dit maintenant movie militer à valeur constitutionnelle et bien que les magistrats puissent progresser et puissent accéder de nouvelles fonctions et tout en respectant aussi leur vie privée parce qu'on sait parfois que notamment pour les femmes, les difficultés pour évoluer sont souvent liées à à cette difficulté de mobilité géographique. Sur l'amendement de notre collègue Lana. Tchétchénie. Alors l'objectif de de notre collègue polynésiennes c'est d'éviter que. Les. Magistrats fassent leur carrière. Uniquement en outre-mer dire d'île en île sans revenir régulièrement sur le territoire métropolitain. C'est pourquoi. Elle inscrit une obligation au bout de 10 ans de revenir de pas avoir une affectation de plus de 10 ans en outre-mer et de revenir pour trois ans minimum en métropole avant à la rigueur de repartir. Nous pensons que c'est une bonne idée. Donc nous sommes favorables à l'amendement de Madame Tchétchénie. Alors Monsieur le Ministre, que vous nous dites-vous, sur l'amendement de Madame Tchétchénie. Ce qu'elle a dit. Madame la présidente, proposer un amendement. La retraite cet amendement. Des le gouvernement. Y sera défavorable je je je veux rappeler que. L'encadrement de la durée d'exercice. Des fonctions et toujours motivée par le souci de protéger l'impartialité dans l'exercice des fonctions partialité encore. Monsieur le sénateur. J'entends évidemment des préoccupations et qui vous conduisent à solliciter l'instauration d'une durée maximale d'exercice des fonctions en outre-mer. Et néanmoins la rédaction vous proposez nécessite d'être retravaillé parce qu'elle vise indistinctement tous les outre-mer. Soit 10 ans d'exercice dans des Outre-mer successifs et non pas au sein du même territoire or imposer un exercice en métropole à des magistrats. Natif d'outre-mer où ils disposent de leurs attaches pourraient être considéré d'une certaine façon comme discriminatoire et je vous propose en conséquence je propose en conséquence que l'on retravaille à une solution qui permette de concilier ces préoccupations et les principes que je viens de rappeler, je suggère donc un retrait de cet amendement est un défaut je l'ai dit j'y serai défavorable. Il en président excusez-moi d'avoir manqué de réactivité. Je n'ai pas eu un réflexe. Suffisamment rapide au regard. Des enjeux de la Polynésie notre collègue là n'Tchétchénie monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, vous l'avez compris. Considère que l'attractivité des fonctions judiciaires est assez différente suivant la nature des Outre-mer concernés et que il y a à l'évidence une appétence plus particulière pour la Polynésie. D'où effectivement des délais d'affectation qui peuvent être importants et qui peuvent être suspendu. Par. Par exemple une nomination. À la Réunion ou autre, ou à une nouvelle Calédonie avant de revenir sur la Polynésie. Ceci étant, vous avez bien compris la nature de la question posée posée par notre collègue je pense que sa logique en évoquant tous les outre-mer était justement de ne pas porter atteinte à l'égalité en ne visant pas spécifiquement la Polynésie mais je prends volontiers acte et j'en rendrai compte à notre collègue que vous êtes ouvert à une réécriture que vous êtes bien conscient qu'il y a quelque part un sujet Polynésie française. Et à cet égard, je pense que notre collègue sera sensible. À ce travail de réécriture, il sera à votre disposition, ainsi qu'à celles de vos services pour travailler en ce sens donc banal président du retrait de l'amendement au regard des explications qu'on nous été présenté. Très bien donc il reste le 69 Corse un avis défavorable de la commission qui est un amendement du gouvernement à métro Woitier pour.

Et il a été retiré, donc il y avait quelque chose peut être d'utile à dire mais il faudra que je le dise autrement. Je ne vous ai pas indûment privé de parole, tout va bien. Donc qui est contre le 69. Bon, il n'est pas adopté et le suivant et. Retiré. Nous avons le 82 de des rapporteurs qui est un amendement de coordination. Si le ministre ne voit pas d'inconvénient à cet amendement et l'Assemblée non plus il est adopté. Nous passons à l'amendement quatre monsieur Cabanel le défend. Oui merci madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues. Cet article donc consiste à à mettre en place les modalités au 3ème quart de pour les magistrats et confie notamment une commission la semaine le soin de dresser arrêter le tableau d'avancement. je vais relayer les observations du Conseil supérieur de la magistrature rendu le 27 avril 2023, il s'interroge notamment sur la légitimité de la commission d'avancement pour procéder à l'inscription au tableau devant du 3ème grade des magistrats il recommande que l'accès au 3e grade soient systématiquement soumis à son approbation. L'objet de cet amendement et donc d'introduire ce mécanisme d'approbation. La commission a rendu un avis défavorable sur l'amendement madame De Lattre. Parce que si on craint ces ces craintes du CSM qu'elle relaye elles sont compréhensibles. Une telle disposition reviendrait à priver la commission d'avancement de l'essentiel de ses prérogatives. Or, elle présente des garanties de représentativité d'indépendance suffisante, donc avis défavorable. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté hein 81 de coordination des rapporteurs, monsieur le ministre, il ne vous pose pas de problème. Il ne pose pas problème. À l'Assemblée les donc adopté et nous passons 61 de madame Vogel. Merci madame la présidente. Donc l'amendement 61, il vise. Élargir le droit de retrouver son son poste pour les magistrats qui prennent un congé parental jusqu'à au moins un an. Vous savez que le congé parental comme nous le connaissons aujourd'hui. Est ouvert enfin donne des droits évidemment. Un salaire et cetera mais aussi à la garantie dans certaines conditions de de retrouver son poste. Sauf que pour les magistrats, les magistrats, la situation est un peu plus compliqué car actuellement. En dehors de cette loi il doivent faire connaître au garde des Sceaux trois choix de réaffectation dans 3 juridictions différentes. À l'issue du congé parental. Ce qui évidemment. Contient beaucoup d'incertitudes, surtout quand on est dans la situation d'avoir un enfant qui vient de naître. Alors le projet de loi apporterait une avancée en garantissant en retour à l'emploi occupé avant le congé parental mais uniquement si le congé parental n'excède pas 6 mois. Or. Les salariés du secteur privé bénéficient d'un congé parental d'un an maximum à l'issue duquel il y peu le feu retrouvé le poste précédemment occupé ou se voir proposer un poste similaire et les fonctionnaires ont le droit de réintégrer leur poste à l'issue du congé parental, indépendamment de sa durée. nous avons simplement cherché avec cet amendement à faire correspondre au moins avec les salariés du privé, le droit pour les magistrats et les magistrats de retrouver leur poste après un congé parental et donc nous poussons la durée de 6 mois à un an. Je vous remercie. Merci. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement. Ça nous comprenons bien évidemment. L'intention de de la rapporteure qui va dans le sens du dispositif bienvenue. Qu'a porté le gouvernement pour permettre effectivement. Plus de transparence dans la gestion des congés parentaux de moins de celui-ci moi et donc de permettre. Aux magistrats de réintégrer leurs fonctions au-delà. Vous proposer d'allonger le délai à un an. Nous, nous pensons que ça risque d'entraîner quand même une désorganisation des juridictions. Donc nous sommes plutôt défavorable à cette mesure de souplesse mais aimerions connaître l'avis du gouvernement sur le sujet. Faut que vous donniez votre avis d'abord. Oui, moi je pense aussi que. Allonger le délai, c'est prendre des risques pour les juridictions. D'autant que d'autant que le magistrat. Après le congé parental peut demander la réintégration dans la juridiction. Vous le savez. Non. C'est une question d'équilibre entre les désirs légitimes évidemment des aide. Des magistrats qui souhaitent prendre congé parental et et la nécessaire prise en compte. Des besoins de juridique des juridictions et là. Je je je me vois contraint de vous dire madame la sénatrice, que je suis défavorable à votre amendement. Madame de La Gontrie, madame la rapporteure maintenant que vous avez entendu l'avis du ministre. Est-ce que ça. Voilà, vous. Madame de la contrition. Sans être totalement étonné je suis consterné de la position du gouvernement parce que ça s'appelle une politique familiale. Donc. On ne cesse de dire qu'il faut encourager à avoir des enfants et cetera et cetera et lorsqu'on veut simplement aligné la situation des magistrats, hommes ou femmes. Aux salariés du secteur privé. Alors là on dit oui mais bon enfin c'est compliqué ouais c'est compliqué parce que c'est compliqué aussi dans le secteur privé. Donc. Il y a quand même un, un sujet. Et le nombre de magistrats est suffisamment important pour que l'on puisse imaginer. Parce que de toute façon si moi ça doit quand même être compliqué aussi, pour les juridictions donc voilà donc moi je je nous alors nous c'est un pluriel de majesté quand. En groupe mais mon groupe. Va soutenir le. si vous savez sous toujours être lucide hein, va soutenir cet amendement très important. Donc je vais mettre aux voix l'amendement 61 madame Vogel, qui a reçu un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté. On dira ce 32 amendements identiques. Le 12. Madame de La Gontrie. Qui consiste à supprimer l'alinéa 172. il est amusant le. L'alinéa prévu dans cet alinéa 172 pour ceux qui veulent. Alors l'idée. Bon on est toujours je pense monsieur le garde des Sceaux en train de chercher des magistrats et donc on s'est dit mais il y a peut-être. Comment on appelle ça, pourvu que ces personnes des seniors. c'est comme ça qu'il faut dire quand on ne veut pas se faire des ennemis. C'est-à-dire aujourd'hui c'est 68 ans, à la limite. Et. Alors il faut dire que c'est un grand succès cette limite d'âge puisque vous savez combien il y a des magistrats qui ont demandé à. Exercer jusqu'à 68 ans trois

Quel est l'avis de la commission. Nous sommes favorables à cette suppression du relèvement de la limite d'âge, on a un vrai objectif c'est ce recrutement de 1500 magistrat. C'est le ministre. C'est une curieuse conception du travail. J'ai j'ai cru que vous alliez dire s'agissant de de magistrats que c'était 2 ans ferme. L'expression qui a été utilisé déjà à moultes reprises me semble-t-il, mais il vous a échappé quelque chose et et ça m'étonne car. Vous êtes toujours en alerte, c'est que c'est sur la base du volontariat.

Bon. Donc je suis défavorable à votre amendement. J'y vois une petite provoque un petit clin d'oeil comme ça bon voilà. Mais pour autant je ne me laisse pas troubler. voulez que je vous dis, puis on va quand même le dire si vous le voulez bien parce que j'ai entendu beaucoup de choses, c'est quand même un métier formidablement passionnant non métier de magistrat comme comme celui d'avocat d'ailleurs. Madame Cohen. Oui, nous voilà rassurés. Monsieur le ministre de la justice. Vous êtes en plein accord avec le ministre du Travail, donc effectivement enfin. Ça concerne, comme l'a dit ma, ma collègue il y a eu trois volontaires, donc là on va légiférer, on va dire mais c'est important et c'est un métier passionnant. Pardonnez-moi, il y a des tas d'autres métiers qui sont passionnants

Monsieur Riché président Richard. Et la limite n'est pas du tout de 70 ans pour ces personnes-là je pense que elle est, elle est à 75 ans et ça permet à beaucoup de de juridiction d'assurer les fonctions d'assurer des missions qu'elles auraient du mal à à soutenir autrement. Monsieur le garde des Sceaux, bien sûr. Je je je veux dire 2 mots là-dessus d'abord d'abord le chiffre de trois je sais pas d'où vous le sortez. Il est contesté. Ben oui moi aussi je vous le dirai mais il est contesté. Bon peu importe, on va se revoir très prochainement donc. Comme on dit nous a fini ben si forcément à se revoir prochainement. ce que mardi je communiquerai chiffre bien. Deuxièmement. Il y a des magistrats à titre temporaire MTT ils veulent servir longtemps leur justice. Notamment quand on va mettre en place l'amiable ils veulent aller assez loin. Hé. Oui 75 ans mais je connais moi plein de. MTT je connais plein de d'avocats qui décident de travailler longtemps et des avocats honoraire d'ailleurs, on les a mis en place. Et des professeurs de médecine et et plein de gens qui n'ont pas envie parce que ils sont passionnés. Non mais OK et quelques sénateurs moi je je je je je ne l'ai pas dit. Mais c'est une mais c'est une réalité, enfin pardon. Non non mais le travail c'est pas voilà c'est 2 ans ferme. Je je sais j'ai compris, moi je suis pas sur cette idée, et je pense que il y a un, ça il y a un certain nombre de magistrats qui seront ravis ravis de servir encore la justice qui les passionne. Bien je vais donc mettre aux voix. Ces amendements qui ont reçu un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient ne sont pas adoptés je mets aux voix l'article 3 qui est pour. Qui est contre. Il est il est adopté. Et je vais faire une petite pause à séance est suspendue, elle sera reprise dans cinq minutes environ. 7.

La séance est reprise et elle est reprise avec l'amendement 15 de madame de La Gontrie. Il est défendu. Oui. Alors comme il est défendu, je demande immédiatement David la. Commission. Dans ces substitution je vous le de critères de difficultés durable de recrutement à celui de difficultés particulières de recrutement. Hé bé écoutez la notion de difficultés particulières de recrutement est déjà utilisée en matière de démographie sanitaire recrutement des fonctionnaires en zone tendue donc cette. Admis et est déjà utilisé en droit constant, donc on prend pas pourquoi il faudrait le changer. Donc c'est un avis défavorable. Je suis désolé. Monsieur le Ministre même avis oui madame la présidente. Je mets aux voix qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté nous passons pardon. Je me vois l'article 4 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté l'amendement 17 madame de La Gontrie, c'est encore vous. Merci madame la présidente. Je souhaite revenir sur certaines modifications qui ont été introduites en commission sur les mécanismes de délégations. En premier lieu. Je suis défavorable à l'élargissement des conditions délégation au profit des cours d'appel, adopté en commission des lois car il ne m'apparaît pas. Répondre aux besoins des juridictions premier c'est de privilégier la première instance et il y a d'ailleurs de très nombreuses lignes qui sont consacrés dans le rapport. Sauvé sur la première instance et il s'agit de concilier tous les impératifs et d'éviter aussi de dévitaliser la première instance. En outre, la procédure d'appel et très spécifique. Peu compatible avec m'dit l'immédiateté et le temps court d'une délégation pour vacances pour un empêchement la même logique vaut pour la fréquence de délégation des magistrats du parquet, il s'agit de dispositifs qui existent depuis plusieurs dizaines d'années et qui ne pose strictement aucune difficulté cet amendement vise donc à revenir à la rédaction d'équilibres antérieurs. Madame la rapporteure. Quel est votre avis sur ces deux amendements. Alors sur l'amendement 17 de madame de La Gontrie. Nous avons un avis défavorable, comme d'ailleurs sur le 70 du Gouvernement sur l'amendement madame de La Gontrie. Donc contrairement à ce qu'évoque les auteurs, il s'agit pas de gérer la pénurie mais pallier d'éventuelles tensions dans certaines juridictions, allez à l'échelle du ressort d'une cour d'appel. Nous sommes opposés au déploiement ponctuel de magistrats de Paris ou d'Aix en Provence qui visait effectivement à gérer la pénurie. Dans le cas d'espèce, il s'agit avant tout d'une faculté de gestion à l'échelle des cours d'appel qui devra effectivement disposer d'effectifs suffisants, nous comptons sur les 5500 nouveaux magistrats. Et nous sommes favorables à une logique de déconcentration, j'y suis particulièrement attaché plus forte à la main des chefs de cour qui seront cette future clé de voûte de l'organisation des concentrés. De la justice en France sur l'amendement 70 du gouvernement. Cette sa rédaction nous paraît beaucoup moins équilibrée que celle. Enfin la rédaction de de la Commission pardon et plus équilibrée que celle du gouvernement. Elle prévoit un équilibre et plus largement les possibilités de délégation à des chefs de cour dotés de moyens de gestion et des ressources humaines renforcé. Ses. Dispositifs de délégations n'ont pas vocation à constituer de mesures de gestion, il apparaît urgent d'en créer plusieurs chefs de cours que nous avons rencontrés pendant des auditions ont déploré l'extrême minceur des leviers de gestion de ressources humaines qui leur sont alloués. Toujours dans cette logique de déconcentration. Et si le gouvernement souhaite évaluer les chefs de cour sur leur capacité de manager de valoriser les fonctions d'encadrement. Ben il importe de leur donner des moyens pour manager justement et encadré. Monsieur le Ministre, quel est votre avis sur l'amendement de Madame de La Gontrie. Bien je vais donc mettre aux voix d'abord le 17 double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté, je me vois de 70 du Gouvernement avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre qui s'abstient n'est pas adopté. Le 16 de madame de La Gontrie est-t-il défendu. Oui. Très bien, que de l'avis de la commission défavorable. Même avis, Monsieur le Ministre. Qui est pour qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 75 du gouvernement. Un amendement laquelle je je je tiens beaucoup. En réalité, il s'agit de ce que l'on a appelé les brigades d'urgence. Qui sont là. Et qui sont composés en cas de crise. De quoi s'agit-il. On demande à des magistrats qui sont en poste qui travaillent déjà. D'accepter pour 6 mois et un jour le un jour correspondant à. Des avantages fiscaux d'aller sur des territoires que l'on qualifie parfois de peu attractif Mayotte Cayenne magistrats et greffiers. On a. Lancé. J'allais dire cet appel d'offres et nous avons obtenu. Très très rapidement. D'innombrables réponse hé bien plus de réponse de magistrats que. Nous avions besoin de magistrats pour composer les dites brigades. Ils sont partis déjà. À Mayotte, les greffiers à Cayenne avec les greffiers et nous avons un un retour d'expérience qui est extrêmement, extrêmement positif. Donc je je je. On avait demandé d'ailleurs puisque nous étions si si j'ose dire hors texte puisque nous le proposons. Dans le texte qui vous est soumis, nous avions proposé au Conseil supérieur de la magistrature. L'autorisation de mettre tout cela en place et le Conseil supérieur de la magistrature. Évidemment a accepté et ces dispositifs de brigade de renfort pour Mayotte et Cayenne. Nous les avons mis en place depuis février 2023, ils ont donné d'excellents résultats sur place. L'avis est unanime. Alors que les tribunaux de Mayotte et de Mamoudzou s'enfoncer dans la crise et avec ces brigades de renfort. Nous avons parer au plus pressé. Il y a dans ces brigades. La notion de crise et ces juridictions mesdames les rapporteurs ont retrouvé un fonctionnement quasi normal nous ont indiqué les chefs de cour et de juridiction. Le mécanisme que je propose est un peu différent mais il aboutit au même résultat renforcer rapidement les juridictions en grande difficulté juridiction d'outre-mer la Corse attends de ce dispositif d'organisation judiciaire c'est pas une mesure de gestion RH. Mais c'est bien un système ponctuel qui vise à éviter une crise. Voilà pourquoi je, j'insiste. Parce que c'est quelque chose qui est récent, c'est quelque chose qui marche bien, nous avons des retours d'expérience qui nous démontre que ça a fonctionné. Mais pourquoi se priver de tels outils. Quelle est la ville la commission sur cet amendement du gouvernement. de faire face à cette surcharge de travail. Nous nous sommes toujours opposés au cédant depuis 2019 à ces mesures qui ne sont que des mesures de gestion temporaire et donc nous restons constants sur le sujet. le garde des Sceaux d'abord les sénateurs après je vous redonnerai la parole si vous êtes d'accord monsieur Merci madame la présidente. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues. Moi aussi lorsque le garde des Sceaux avait. Annoncé ces brigades. J'étais sceptique. Ce sont des sujets que je suis de près parce que dans nos territoires en difficulté. Si en plus la justice dysfonctionne. La la population. Bien sûr. Et comme vient de le dire le le garde des Sceaux. C'est une satisfaction mais total et unanime, je suis très en lien avec les auxiliaires de justice, que ce soit les avocats ou. Les les huissiers de justice. Et c'est vrai qu'au départ, tout le monde était un peu circonspect mais force est de constater que ces brigades ponctuelles viennent. Pour le moment soulagé les les les tribunaux en commençant par écumer les énormes retards. Alors c'est vrai, ce n'est pas une solution pérenne. Je suis le 1er à ne pas le souhaiter, mais force est de constater que cet apport ponctuel et utile et tant que. L'attractivité effectivement de nos territoires ne sera pas revenue. Nous avons besoin. De, de ces, de ces brigades et c'est pour ça que vraiment cher collègue. Je comprends les réticences de mesdames les les les rapporteurs, elles sont légitimes. Mais c'est quelque chose qui marche. Qui n'a pas vocation à se pérenniser. Mais en attendant, nous en avons extrêmement besoin et c'est pour ça que j'insiste pour que. Nous adoptions cet amendement.

Une rustine. Emplâtre sur une jambe de bois, mais pas du tout. On règle la l'urgence. La crise au réuni très, très vite on en voit très vite six mois. Et puis ensuite. Les choses. Naturellement une fois que les Brigades ont fait leur action et elles font leur action mais. Ça ça ça n'est pas en contradiction avec ce que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire. Améliorer l'attractivité l'attractivité, elle s'améliore, avec des rémunérations. Elle s'améliore aussi avec un système que nous mettons en place. Système de mobilité. Vous en avez parlé. C'est-à-dire qu'un jeune qui acceptent d'aller là-bas à Mamoudzou, pardon de le dire, il y a pas. Une salle de spectacle. Il y a de l'insécurité. C'est terriblement difficile, il faut avoir envie d'y aller. On a mis en place d'ailleurs des billets d'avion je je je vous livrent cette anecdote mais elle est significative des difficultés pour permettre à des jeunes qui sont jeunes et qui ont 20. 20 et quelques années de pouvoir aller de temps en temps sur l'île de la Réunion pour passer un week-end normal j'allais dire Et sur les questions de mobilité. Ce que l'on fait c'est que ceux qui acceptent d'aller là-bas on leur garantit quand leur mission est terminée, un poste qu'ils auront choisi qu'ils ont près choisi si j'ose dire. Donc oui c'est pas en contradiction avec ce que nous faisons pour davantage d'attractivité. C'est une notion de crise et d'urgence. Et moi je pense que en cas de crise et d'urgence. On a été en réalité très heureux d'avoir trouvé système on a été ravi de mettre en place et je peux dire que tout l'écosystème s'est félicité de cela. Alors moi je je je je pense que au-delà de des choses qui peuvent nous opposer des visions qui peuvent être divergentes. Puis c'est bien le moins dans une dans une grande démocratie et dans un débat parlementaire mais enfin ça ça marche et ça fonctionne et il ne s'agit pas pour la chancellerie de dire on a mis ça en place on

C'est parfaitement de quoi je parle et et et de l'efficacité de l'efficience de ces brigades d'urgence à Mayotte. On en avait tellement besoin. Donc ne nous privons pas de ce dispositif, il a pas vocation ce dispositif à à boucher les trous c'est c'est pas ça l'histoire je je je l'ai dit, mais dans l'urgence on peut composer très vite des brigades et ces brigades ont une véritable utilité. C'est un outil nouveau c'est pas du tout pour remplacer, je ne sais quoi, c'est pour créer quelque chose qui permettent de faire face à une situation de grande crise. Voilà le dispositif et, et voilà pourquoi je je me permet de redire ici que je suis fondamentalement attaché à ce dispositif. Oui. Nous attendons effectivement il y a 2 sujets il y a le sujet de fond c'est de rendre plus attractif. Ces postes en Outre-mer ou même en Corse, qui même si je trouve que l'association des deux paraît parfois surprenantes pour rendre plus attractif ces ces néanmoins nous il y a plusieurs choses, d'une part. La crise et les crises dans les juridictions, elles existent aussi en métropole et on a trouvé des solutions et déjà vous avez trouver des des solutions. Pour répondre aux crises dans l'urgence, là c'est. Quand même vous inscrivez de manière pérenne dans un projet de loi organique, je le rappelle tout de même. Un dispositif qui vise à répondre à des situations de crise alors que nous, nous pensons que il faut au maximum éviter ces crises en créant des moyens supplémentaires et pourquoi pas en mettront temporairement des moyens via les sucres rapides via d'autres systèmes et donc là vous vous voulez pérenniser dans le PJ Un dispositif qui vise à répondre à des situations de crise. Prenant acte et maintenant ces dispositions comme en fait. Je ne veux pas éternisée cet. Cet échange mais d'abord les sucres rapides ne sont pas des magistrats. Premièrement. Non mais d'accord, ce ne sont pas des magistrats. puis deuxièmement, c'est sur la base du volontariat. Certes on inscrit dans la loi organique. Mais c'est sur la base du volontariat, on ne force pas des gens à aller. Le problème, vous me dites mais. Au fond ce que vous dites, vous dites, bon très bien puisqu'on a les moyens on va embaucher davantage de magistrats, on va régler la question mais non. Pas forcément. Pas forcément parce que il faut les trouver les magistrats et les greffiers qui acceptent. Ces territoires dont on dit parfois qu'ils sont. Difficiles et ils le sont. Donc. La réduction si vous voulez du du du temps ces six mois ça incite évidemment un certain nombre de de jeunes magistrat c'est plutôt le profil sont de jeunes magistrats. Aller là-bas et et et à régler les difficultés. C'est pas encore une fois c'est pas la règle commune qu'on met en place là. C'est un dispositif qui sert. Kant, on est vraiment en Bolliger Kant, on n'arrive plus à rendre la justice. Bien je vais donc mettre aux voix cet amendement du gouvernement qui a reçu un avis défavorable de la commission qui est pour. Qui est contre ou qui s'abstient. Il n'est pas adopté l'article 5 qui est pour. Qui est contre qui. Ça se tient. Il est adopté à l'article 6, madame.

Donc le 21, quel est l'avis de Madame rien défavorable. Monsieur le Ministre même avis. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient pas adopté le 18. Madame de La Gontrie. Défendu. Voilà défavorable. Voilà monsieur le ministre aussi de la tout. Mais surprenez-nous. Donc il est. Même vote que le précédent, donc il n'est pas adopté le 19. Madame de La Gontrie.

Pour éviter un émiettement syndical. Sauf que, aujourd'hui, le seuil est à 6%. Donc vous allez favoriser un peu plus l'émiettement syndical donc défavorable. Vous le retirer. Vous le maintenez l'avis du gouvernement, le même.

Défendu. Des défavorable. Monsieur le ministre aussi. Même vote que sur le précédent l'article 6 ce qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'article 7. Nous avons un amendement 66 de Monsieur Mohamed Soihili. Le précédent n'étant pas défendu. Oui madame la présidente, très rapidement. Cet amendement vise à préciser les attributions que les magistrats exerçant à titre temporaire, les fameux. MTT dans les fonctions de substitut peuvent se voir confier ses attributions sont saines du ministère public de les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police et en matière de mise en, en oeuvre des alternatives aux poursuites et d'ordonnance pénale. Par ailleurs, nous proposons de supprimer la disposition adoptée par la Commission visant à interdire la participation de MTT au jury professionnel. Cette disposition en effet est déjà prévue par les textes, relatifs au jury professionnel. Merci. Quel est l'avis de la commission. C'est une propose c'est une proposition qui semble. Effectivement bienvenue une sagesse positive. Monsieur le Ministre. Je suis favorable. Madame la présidente. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis de sagesse de la commission et un avis favorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté l'article 7 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'article 8, nous avons un amendement 26 madame de La Gontrie. Nous demandons simplement l'application de la loi Sauvadet. Qui qui édicte une obligation de 40% de chaque sexe pour les nominations dans les emplois supérieurs de l'État. Quelle est la ville la commission. oui et je pense que par contre, je suis tout à fait d'accord sur le principe le le problème semble-t-il aujourd'hui et donc qui mérite d'être. Monsieur le ministre, hein. Donc le problème, ce serait qu'imposer un quota pourrait. Faire l'objet d'une mise en oeuvre complexe compte tenu du rôle que tient le Conseil supérieur de la magistrature de la nomination à ce poste mais ah sociaux le à la démarche de réflexion. ça pourrait aussi avoir une difficulté constitutionnelle au regard des principes Naveau Billy d'inamovibilité et d'égalité de traitement, donc une transposition pure et simple des dispositions applicables aux fonctionnaires introduite par la loi Sauvadet dans leur donnant statutaire a été écartée. vous donnons donc un avis défavorable mais à titre personnel, je vous invite. Monsieur le garde des Sceaux a travaillé sur ce sujet. Monsieur le garde des Sceaux. Je vais travailler, madame. La rapporteure. Défavorable. Donc je mets aux voix cet amendement, qui assume qui a reçu un double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 41 monsieur Bonnecarrere. Oui madame. Le président, mes chers collègues. L'article 41 pose la question de la négligence. Ce qui y être une question qui fait bien sûr et réagir immédiatement. Les syndicats de magistrats. disons-le immédiatement. Notre groupe est modérés particulièrement a le sens des responsabilités. Nous comprenons bien la crainte des magistrats d'être mis en cause personnellement. Entre cette crainte. Et la situation que chacun de nous connaît. Où il n'y a aucune mise en cause il y a probablement place. Pour des solutions intermédiaires. La question que nous posons. Et la question. Finalement de l'insuffisance professionnelle qui existe dans tous les métiers, elle exige les avocats. Elle existe dans toute l'émission là existe donc aussi chez les parlementaires et elle peut aussi exister chez les magistrats. Je comprends demande bien dans la réaction du ou des syndicats de magistrats. Que l'on souhaite que cette notion de négligence ou cette notion d'insuffisance professionnelle soit mieux appréhender mais elle ne peut pas être écarté de notre regard et notre. J'ai quartier immédiatement 2 arguments l'qui consisterait à dire, si vous me parlez de négligences qui doit par ailleurs correspondent à des violations répétées et caetera, il faudrait un sujet d'assurance non on est bien dans une responsabilité et on ne va pas mélanger la question des des élus dans un parallèle pénal disciplinaire. Il y a bien longtemps que la responsabilité des élus, prend en compte la nature l'émission des fonctions des compétences des moyens dont on dispose, c'est-à-dire l'idée d'une appréciation in in concrète au il n'est nullement mon entrée mention d'avoir un régime plus favorable pour les élus que pour les magistrats. Donc monsieur le garde des Sceaux. Nous serons attentifs, comme nous l'avons été sur autre observation concernant tout à l'heure la notion d'impartialité a travaillé sur une rédaction la plus qualitatif possible mais on ne peut pas écarté d'une pichenette. La notion de négligence et derrière la question de l'insuffisance professionnelle. Merci. Quel est l'avis de la commission sur cet amendement. Favorable. Madame la présidente. Gouvernement. Merci madame la présidente, monsieur le sénateur Bonnecarrere. Je partage. Votre avis selon lequel le régime disciplinaire des magistrats doit être renforcée. C'est d'ailleurs le sens du texte que j'ai présenté à votre assemblée. Pour autant. Le régime de responsabilité des magistrats. Obéit. Comment le dire de subtils équilibres constitutionnels. Le 1er mars 2007. Le Conseil constitutionnel le rappel d'ailleurs clairement. Si les principes d'indépendance de l'autorité judiciaire. Et de séparation des pouvoirs n'interdisent pas au législateur. D'étendre la responsabilité des magistrats. À leur activité juridictionnelle c'est je cite. À la condition. Que l'engagement de poursuites disciplinaires. Repose sur une violation des des devoirs de son office préalablement constaté par une décision de justice. Il me semble qu'en l'état de votre rédaction. La définition de la faute que vous proposez. Ne. Comprend pas les garde-fous exigés par le Conseil constitutionnel. Et risque ainsi d'être censuré. Il ne faut pas omettre que les magistrats apprécient souverainement. Souvent de façon collégiale. Les faits qui leur sont soumis. Il en va de même pour l'introduction de la notion de négligence qui risquerait bien sûr d'être considéré comme excessivement flous. Et de plus, cette disposition n'apparaît pas forcément utile. Pourquoi. La jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil d'État est clair. L'erreur d'appréciation. Ou d'interprétation ne saurait constituer une faute disciplinaire. En revanche. Il est aujourd'hui parfaitement possible. De rechercher la responsabilité du magistrat à raison d'un acte juridictionnel. Dès lors que l'acte est détachable de l'activité juridictionnelle. Le CSM. A également sanctionner des magistrats en cas de négligence multiple. Je pense par exemple à une affaire jugée en 2022 dans laquelle un juge d'instruction a été sanctionné pour de multiples retards des négligences dans le traitement de ces dossiers ayant donné lieu à des remises en liberté ou encore une autre affaire ou une juge a été sanctionné pour des retards dans le rendu de ses délibéré enfin. La protection de l'acte juridictionnel n'est pas garanti. Qu'au niveau national mais également et vous le savez au niveau européen pour toutes ces raisons et à la lumière des précisions que je viens de vous apporter. Je suggère à ce stade, un retrait de votre amendement.

Je retire même si la question de la négligence doit bien être à mon avis restait posée. Très bien. Nous passons à l'amendement 32 de madame de La Gontrie. Cet amendement. Profite du du du projet de loi qui nous est présenté pour. Proposer une refonte globale du régime des sanctions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire. Est ainsi proposé 4 groupes de manière à mieux les hiérarchiser. D'une part. En fixant les règles relatives à l'effacement des sanctions du dossier. En fonction du groupe auquel ces sanctions appartiennent et d'autre part avec le prononcé d'une sanction du deuxième ou troisième groupe pendant une période de 5 ans après le prononcé d'une exclusion temporaire. Cela entraînerait la révocation du sursis et enfin l'instauration d'une mesure infra-disciplinaire qui serait un rappel au devoir et qui serait en encadrée de la même manière. Vous voulez présenter le 25 en même temps en fait. J'allais vous le proposer. Le 25 propose de supprimer l'allongement de la durée qui est prévu dans le projet de loi de l'inscription des avertissements dossier des magistrats. Précisons que l'inscription des avertissements à ses dossiers et d'ores et déjà une mesure dérogatoire. Ni le code général de la fonction publique, ni le code de justice administrative ne prévoit l'inscription des avertissements aux dossiers des fonctionnaires. Et. Aujourd'hui, alors même que cette durée de trois ans, vous proposez de la passer à 5 ans, cela nous semble excessif et donc nous voulons supprimer. Il suffirait. Madame. La présidente a ceci est ce coup dur présenter l'identique à celui de Madame de la gauche. Mais je veux dire simplement 3 lignes quand même. je vous ai demandé de présenter. Oui, dans cette simplement pour expliquer pourquoi vous nous voulons supprimer cet alinéa, tout simplement parce que pour. Cette suppression donc vise à garantir selon nous une équité de traitement entre les magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif et donc nous voulons ici souligner que l'inscription des avertissements au dossier et déjà une mesure exceptionnelle pour les magistrats de l'ordre judiciaire et un délai de 3 ans selon nous également offre amplement le temps nécessaire pour évaluer et prendre en compte les avertissements reçus. mesdames les sénatrices messieurs les sénateurs, je je partage évidemment la volonté, je l'ai dit déjà. Du renforcement du régime disciplinaire des magistrats. Mises en Oeuvres par le texte de la commission. Mais. Certaines incohérences me semble devoir être corrigée. Par le biais du présent amendement. Qui peut concevoir qu'un magistrat qui n'exerce plus les fonctions de juge d'instruction. Se voit retirer ces mêmes fonctions. Même si les manquements pour lequel il est sanctionné ont été commis alors qu'il exerçait cette fonction de magistrat instructeur prononcé cette sanction vous me le concevrais n'est pas possible et n'a pas de sens de même. Je ne vois pas la raison pour laquelle l'ordonnance statutaire devrait être alourdie de texte qui vise les fonctions spécialisées l'interdiction d'être nommé juge unique recouvre déjà et évidemment toutes les fonctions spécialisées vous ne pourrait pas être nommé juge des enfants, juge de l'application des peines, juge d'instruction JLD. Si une telle sanction. Vous êtes infligé car il s'agit de fonctions qui s'exerce seul. Si vous êtes nommé juge non spécialisés. Le président pour vous désignez ne pourra vous désignez que pour exercer dans des formations collégiales. C'est le sens de cette sanction n'est pas utile, à mon avis de préciser les différentes fonctions qui sont concernés. Je suis favorable en revanche à la redéfinition des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire et je vous présente cet amendement afin que cette échelle des sanctions soit efficiente et efficace. C'est l'efficacité de la procédure disciplinaire qui me guide également à présenter une proposition d'allongement du délai dans lequel le conseil de discipline doit se prononcer sur une interdiction temporaire d'exercice. Cette mesure n'est pas une sanction, c'est une mesure probatoire qui répond à l'urgence, elle est prononcée. Lorsque l'intérêt du service public de la justice commande que le magistrat souhaite immédiatement sorti du tribunal dans lequel il exerce cette mesure est donc grave elle nécessite que le garde des Sceaux, ministre de la justice. Dispose d'un délai suffisant pour rassembler les pièces, appuyant sa demande mais surtout que le magistrat bénéficient d'un délai suffisant pour préparer sa défense, ce sont ces raisons qui m'ont convaincu de présenter l'amendement. Madame la rapporteure. Quel est votre avis sur ces amendements alors. Tout d'abord sur le 32. De. De madame de La Gontrie qui propose une refonte de l'échelle des sanctions sur le modèle applicable aux magistrats administratifs, nous avons pris en partie et effectivement modèle mais pas totalement sur les magistrats administratifs, donc cet amendement, nous semble un peu excessif. C'est pourquoi nous émettrons un avis défavorable. Sur d'ailleurs nous nous tu sont sommes tenus au conseil du CSM sur les amendements, 25 et 48 de madame de La Gontrie et de Madame Cukierman enfin du groupe communiste. Nous sommes défavorables à l'évolution proposée portée de 3 à 5 ans l'inscription de l'avertissement dans le dossier du magistrat est aussi une recommandation du CSM de son avis du 24 septembre 2021. Côte à l'amendement du gouvernement. Alors nous notons. Monsieur le Ministre, l'avancée que vous faites vers nous pour autant vous nous retirer beaucoup. De nos préconisations qui sont nous l'entendons probablement imparfaite et mériterait d'être. Nous avons la navette donc nous mettons pour l'instant un avis défavorable à votre amendement mais somme tout à fait conscient qu'il y a à retravailler sur le sujet. Il n'y a pas d'explication de Monsieur le Ministre, c'est à vous. D'autres amendements. Si madame la présidente. Je suis défavorable à l'amendement 32 comme je suis défavorable aux amendements, 25 et 48. Quant au travail. Ça me fait pas peur. Le travail, donc on va travailler ensemble. Pour améliorer ces dispositions. Donc je aux voix d'abord le 32 double avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Le 25. 48 même vote même vote le 67 du gouvernement avec avis défavorable de la commission qui est pour. Qui contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Nous passons à l'amendement 27 madame de La Gontrie. Il est défendu. Quel est l'avis de la commission. Défavorable l'avis du Gouvernement défavorable. Qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. Il n'est pas adopté le 31. Madame de La Gontrie. Merci madame la présidente. Nous voulons introduire de garanties procédurales essentielles devant la commission d'admission des requêtes aujourd'hui une décision d'irrecevabilité ne fait l'objet d'aucune obligation d'information, c'est un petit peu curieux. Donc nous proposons que une plainte déclarée irrecevable. Que que lorsqu'une plainte est déclarée recevable. Son auteur en soit informé. Mais par ailleurs, nous proposons également que lorsque la plainte est recevable. La commission et pour. Obligation de la transmettre magistrats concernés alors qu'aujourd'hui la la seule obligation d'en informer de l'informer de l'existence mais pas de lui transmettre la plainte. Voilà les 2 améliorations de procédure que nous proposons. Devant la commission des requêtes. déjà que le magistrat visé par la plainte le justiciable chefs de cour visé au 9ème alinéa du présent article sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire, ce qui ne remet pas en cause l'article 8 l'alinéa 8 du même article 51 trois prévoit déjà que le magistrat est informé d'une éventuelle recevabilité. Il ne semble donc pas que la communication de la décision soit d'une pertinence particulière à la suite de la procédure soit qu'elle soit rejetée, soit qu'elle donne lieu à une poursuite d'ici. CCleaner, donc avis défavorable je mets aux voix. Monsieur le Ministre par donc

du rejet d'une plainte contre un magistrat ou s'il y a lieu de l'engagement d'une procédure disciplinaire. Le projet de loi prévoit d'aller au-delà de cette simple et nécessaire, obligation d'information. Apparemment monsieur le garde des Sceaux, vous souhaitez obtenir le droit de demander à la commission d'enquête des requêtes je cite toutes pièces de la procédure. Si j'ai bien compris toutes pièces de la procédure. Ça signifie. Potentiellement les notes. Et Toutes les pièces qui auront lieu à la procédure sachant que peut-être que cette procédure dont n'aura pas lieu. Effectivement à l'ouverture d'une enquête comme. Le ministre de la justice n'est pas responsable du contrôle de la recevabilité des plaintes et n'a pas besoin d'avoir accès à tous ces détails. J'avoue que nous ne comprenons pas trop pourquoi. Ça vous paraît nécessaire. Nous proposons de le supprimer et à la limite. Si j'imagine comme c'est le cas, vous y êtes défavorables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous considérez qu'il est juste nécessaire et proportionnée, que le garde des Sceaux et accès à toutes les pièces de la procédure, y compris lorsque des magistrats ne vont pas être ensuite mis en cause.

oui oui oui tout ce excusez moi c'est rien. Donc. Ce sont des avis alors pour tout ce qui est la suppression de la communication, garde des Sceaux des décisions est recevable. Ce sont des avis défavorables La transmission des plaintes jugées recevables doit permettre au garde des Sceaux la phase pré-disciplinaire étant closes d'examiner l'opportunité de poursuivre d'éventuelles fautes disciplinaires qui seraient susceptibles, usant de ses prérogatives diligenté une une enquête administrative par exemple d'engager.

Il est effectivement utile que si la car. Décèle une des difficultés déontologique dans l'examen de la plainte de justiciables elle puissent relayer cette difficulté et faire ainsi fructifier les travaux qu'elle a conduit. deuxièmement, cet amendement semble. Permet de contourner une une éventuelle difficulté constitution nel. Si la carte pourrait difficilement au regard des attributions du CSM procéder elles-mêmes un rappel des obligations déontologiques. Il est néanmoins utile que des éléments d'information soit transmis aux chefs de cour qui pourra lui exercer ses attributions en la matière. Merci madame la présidente suisse défavorable aux amendements. 29 49. 64. S'agissant de l'amendement déposé par Madame Vogel. Peut le garde des Sceaux une compétence en matière disciplinaire. Et il est normal que le garde des Sceaux veuille être le plus parfaitement possible éclairé par là. Ça me paraît d'ailleurs une bonne mesure et. Et une garantie que le garde des Sceaux est taxé. Aux éléments du dossier avant de prendre quelque décision. Que ce soit ça devrait pleinement vous vous rassurer. Non je suis défavorable à ces amendements. En revanche, je suis favorable à l'amendement de monsieur sénateur Bonnecarrere. Transmission de l'ensemble des décisions de la aux chefs de cour. Ça me paraît une bonne mesure. Alors je vais donc mettre aux voix d'abord le 29 autour de l'avis défavorable qui est pour. Qui est contre qui s'abstiennent n'est pas adopté même vote sur le 49, j'imagine. Je mets aux voix le 39 double avis favorable qui est pour. Qui contre qui s'abstient il est adopté et le 64 même votre que sur le 29. Il n'est pas adopté 2 amendements en discussion commune. Nous commençons par le 28 de madame de La Gontrie. Défendu.

Non j'ai dit défavorable à à celui de madame de La Gontrie. Est favorable à celui de Monsieur Bonnecarrere. Pour monsieur le garde des Sceaux même. Avis ou non. Dites-moi Pardon. Ah vous m'entendiez pas. Lever toute ambiguïté, je suis défavorable à l'amendement que vous avez déposé. Quant à l'amendement qui est déposé par Monsieur le Sénateur. Bonnecarrere, je vais faire quelques remarques. Je suis. Opposé Monsieur le Sénateur au changement de de de paradigme que vous proposez. Parce que si la demande d'enquête administrative, rejeté par le garde des Sceaux. Il reviendra à la Car ou au rapporteur. Ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire d'en tirer toutes les conséquences sur les éléments dont il dispose. Pour apprécier la situation qui leur est soumise, et il leur reviendra également de l'évoquer à l'audience à laquelle un représentant du garde des Sceaux est présent. D'autre part. Et surtout. Il convient de rappeler que l'inspection générale de la justice et placée sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice. Et transformer le silence de ce dernier. Dans un laps de temps très contraint. En décision implicite d'acceptation reviendrait en réalité à priver le garde des Sceaux de son pouvoir d'appréciation de saisir l'Inspection aux fins aux fins d'enquêtes administratives et vous comprendrez dès lors que pour l'ensemble de ces raisons. Ma position est défavorable. qui compte qui s'abstiennent n'est pas adopté le 40 avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement qui est pour. Qui est contre on qui s'abstient. Il est adopté. Le 63, madame Vogel. Il est défendu, je crois. Et quel est l'avis de la commission sur l'63 défavorable avis du gouvernement. Même avis défavorable. Monsieur le Ministre sur l'A 63 ou peu. Oui. Oui c'est défavorable. 63. Je ne peux pas trop le supposé non plus vous savez. Donc je mais on voit. Qu'il est pour. Qui est contre qui s'abstiennent n'est pas adopté l'article 8 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient-il être adopté après l'article 8. Madame Boyer de 58. Merci beaucoup madame la présidente. J'ai l'honneur de défendre ce cet amendement qui a été présenté par le président Retailleau est cosigné par bon nombre de nos collègues. dans l'esprit des états généraux de la justice le président Retailleau a souhaité en complément de la redéfinition de la faute disciplinaire qu'on s'attarde sur la faute déontologique et que pour que les Français qui nous écoutent, comprennent. Je voudrais rappeler qu'il y a la faute disciplinaire dont on vient de parler, mais aussi la faute déontologique. C'est pourquoi le présent amendement entend créer une charte de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire à l'instar de celle qui a été élaboré à destination des magistrats de l'ordre administratif. En vertu de la loi d'avril 2016 qui est relative à la déontologie, au droit des obligations des fonctionnaires. C'est pourquoi le président Retailleau souhaite modifier l'article 20 de la loi organique de. Février 94 sur le Conseil supérieur de la magistrature qui confie à ce conseil, je le cite le soin d'élaborer et de rendre public un recueil des d'obligations déontologiques des magistrats. L'emploi du terme recueil traduit l'ambiguïté de la portée de ces dispositions. En effet, la charte de déontologie des magistrats administratifs, constitue un écrit solennel engageant et complet, et non un simple catalogue de recommandations telles qu'il existe actuellement pour les magistrats judiciaires en outre l'amendement associés à l'élaboration de cette charte de déontologie. Les instances les mieux à même de définir avec précision les règles déontologiques applicables aux magistrats judiciaires. Le directeur général de l'administration de la fonction publique, la commission de déontologie de la fonction publique. Le collège de déontologie des magistrats de leur judiciaire l'inspection générale de la justice, ainsi que les organisations syndicales représentatives de la magistrature. Et donc je j'espère que vous conviendrez que cet amendement peut recueillir en tout cas je je le souhaite et je crois que nous l'espérons tous l'assentiment de l'ensemble de cet hémicycle. Quel est l'avis de la commission. Favorable. Madame la présidente. Il nous semble effectivement qu'une charte. Serait plus engageante qu'un recueil. Et les consultations prévues sont de nature à favoriser l'acceptabilité de cette charte. Donc favorable. Monsieur le Ministre. Je suis également favorable. Madame la sénatrice mais. Ne vous réjouissez pas trop vite et toute petite réserve m'expliquer. Aujourd'hui voilà ce que nous avons nous avons. Un recueil des obligations déontologiques des magistrats. Je trouve que. L'idée que vous développez qui est porté par le président Retailleau est une idée intéressante et qu'elle était opportune. Je le dis sans ambages. La charte permettra de clarifier les obligations déontologiques des magistrats. Et de les fixer. À l'instar, vous l'avez rappelé le ce qui existe déjà pour les juges administratifs. Je m'interroge simplement sur la consultation du directeur général de la fonction publique et de la Commission déontologie de la fonction publique dans la mesure où les magistrats de l'ordre judiciaire. Ne sont pas des fonctionnaires. Donc là il faut que l'on fasse très très attention. Et en outre le système de consultation que vous proposez. Va nécessiter de modifier les attributions du collège de déontologie. Limitativement énumérées à l'article 10 tiré de du statut de la magistrature et ne renvoie pas à un tel avis. Alors pour les mêmes raisons. Nous devons prévoir de redéfinir les attributions de l'inspection générale de la justice. Donc. Oui sur le principe. Je souhaite que on poursuive le travail dans le cadre de la navette. Et je suis évidemment. Favorable. À l'amendement. Sous les réserves que je viens. D'exprimer, nous avons le temps de retravailler. Cet amendement et de bâtir ensemble. Cette charte. Madame de La Gontrie pour l'explication de vote. Décidément. Évidemment une charge supplémentaire contre. La liberté d'expression, la liberté syndicale les obligations des magistrats. L'occasion était trop belle. Je dis cela parce que. Très peu d'amendements du groupe LR dans son ensemble notamment du président Retailleau. Je crois qu'il y en a eu deux vous trois, dont un d'ailleurs qui a été rejetée par le Sénat. Mais voilà une charte de déontologie. Alors le le le président Retailleau il. quand il s'attaque aux magistrats, il ne va pas avec le dos de la cuillère comme on dit. Début du mois de mai. Il dit. Il y a un problème avec le CSM. Qui est totalement corporatiste. Il faut des sanctions contre le syndicat de la magistrature. Et il n'exclut pas. L'idée de travailler sur l'interdiction de de de du droit de se syndiquer. Pour les magistrats. Vieille rengaine de la droite. Donc. Sans doute. Consultant un certain nombre de. Documents et de de droit constitutionnel et s'est dit que c'était quand même peut être un peu compliqué. Alors on a déjà le garde des sceaux qui lui sert sur un plateau. Une saisine du Conseil super la magistrature. C'est d'ailleurs exactement aux mêmes dates.

Je pense que nous serons toujours opposés à ce type de démarche et la Charte de temps le dos logis n'est qu'un faux-nez de cette démarche là. Très bien je vous remercie. A-t-il d'autres explications de vote, monsieur le garde des Sceaux. Pour une intervention. À. Oui très rapide, je vous rassure. Faut pas voir le mal partout et le fantasme. On ne peut pas tenir lieu de de raisonnement, me semble-t-il. Ce texte. Il est là je je l'ai pas inventé pour les besoins de la démonstration. Il précise un certain nombre de choses, j'en ai lu un extrait tout à l'heure sur l'obligation de réserve par exemple bon. Qu'est-ce qu'il y a de mal pardon mais. A demandé au Conseil supérieur de la magistrature son avis. Moi j'aimerais comprendre si je l'avais fait d'autorité, alors là vous pousse charrié des cris d'orfraie en disant je je ne sais quoi, enfin je vois à peu près quoi. D'ailleurs, mais là il s'avère que je demande qu'on si je gouverne à la magistrature de Monsieur le Sénateur. Bonnecarrere présente son amendement. Je dis attendons son avis très respectueux. J'ai dit tout à l'heure que pour l'évaluation des chefs de cour, j'ai demandé au Conseil supérieur de la magistrature que je veux voir régulièrement et son avis m'importe mais est-ce que des magistrats dans leur expression individuelle ou dans leur expression syndicale ont quelque chose à craindre du Conseil supérieur de la magistrature. Faut être sérieux pas toujours la peine de sortir. Je ne sais qu'elle qu'démon là. Pour faire dire le le le contraire de ce que souhaite moi je pense qu'une charte, c'est plus clair. Pas plus compliqué que ça et j'ajoute. Si vous le voulez bien. Que pour la construction ces chartes naturellement il faut également qu'on demande l'avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ça me paraît une évidence. Voilà. Conseil supérieur de la magistrature. Vous savez. Ah déjà rendu au président de la République. Un rapport sur la responsabilité des magistrats. Et il est allé bien plus loin que ce que l'on faisait autrefois Conseil de supérieur de la magistrature a conscience d'un certain nombre de gens, il ne faut pas tout voir sous sous l'angle et et à l'eau de je sais quelle volonté de vous voyez, ça n'est pas comme ça que les choses se passent. Voilà moi l'expression syndicale. Je vais vous dire, madame. La sénatrice. Je l'entends je la regarde et je ne la commande pas. Et la Et la liberté syndicale. Elle existe, elle doit être garantie dans notre pays. Et je pense pouvoir dire qu'elle est. Madame Boyer pour une explication de vote. Il sera très intéressant effectivement d'améliorer cet amendement et de le peaufiner, dans le cadre de la navette parlementaire c'est sûr mais je voudrais simplement vous rappeler que nous, nous avons été nombreux à participer aux états généraux de la justice et je pense qu'un tel amendement est aussi issu de ces travaux est propre à réconcilier. Les Français avec la justice et que une charte bien c'est quelque chose qui est consultable qui est clair, qui est élaboré en commun et qui permettra probablement d'améliorer les choses. C'est la raison pour laquelle le président Retailleau a présenté cet amendement que nous avons été nombreux à le soutenir et que j'espère nous allons le voter. Je vous remercie. Bien si les obligations de vote ont terminé je suis saisie sur cet amendement 58 de de demande de scrutin public une du groupe LR et une du groupe socialiste, écologiste et républicain. Je rappelle que l'avis de la commission est favorable que l'avis du gouvernement est favorable et que le scrutin est ouvert.

Personne ne demande à voter

Bien plus personne ne demande à voter le scrutin est clos. Et sur cet amendement 331 votants exprimés, 317 pour 298 et. Contre 79. Le Sénat a donc adopté, je me vois l'article 9 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient il est adopté à l'article 10. Madame de La Gontrie défendu. L'amendement 24. Oui. D'accord que les l'avis de la commission sur ces amendements. En fait. Pour moi il il est satisfait puisque depuis l'entrée en vigueur du RGPD n'est plus nécessaire de passer par un tel décret comme celui qui. Je voulais te demander donc défavorable.

hé bien voilà Monsieur Vial, allez. L'amendement. Merci madame la présidente. C'est un amendement qui est présenté par mon collègue et notre collègue Max Brisson. Afin de de supprimer cet article 11 qui prévoit l'expérimentation d'un concours spécial destiné au recrutement d'étudiants issus des des prépas talent titulaire a minima d'un bac et boursiers en 1er lieu, il convient de rappeler que l'École nationale de la magistrature l'ENM a ouvert ces dernières années des classes préparatoires ces pays aujourd'hui au nombre de dans le pays, pouvant accueillir jusqu'à 108 préparation nerfs ces préparations gratuites sont destinées aux étudiants boursiers méritants qui souhaitent préparer le 1er concours d'accès à la magistrature le concours dit étudiant. Dès lors, les auteurs du présent amendement ne perçoivent pas l'utilité d'expérimenter un concours différents alors que ces préparations nerfs ont déjà vocation à préparer le concours commun l'ensemble des étudiants et deuxièmement si on ne peut s'opposer par principe aux solutions de toute nature permettant de favoriser la diversité du recrutement dans la magistrature. Le niveau de compétence attendu doit être le même pour tous, ça ne semble une question aussi de justice la l'instauration d'un tel concours spécial ne sommes donc pas satisfaisant pour le corps judiciaire. Nous proposons donc la suppression de cet article. Très bien qu'elle est la ville la commission sur cet amendement. encore plus l'accès à la magistrature auquel nous sommes attachés et elle s'accompagne déjà de garantie bienvenue et elle est à l'image de ce qui existe déjà pour l'accès. Despé. Donc nous pensons que c'est une bonne solution c'est prépa talent, donc nous sommes contre leur suppression. Monsieur le Ministre. Je suis très attaché à l'ouverture et très attachés à l'ouverture sociale. Ça me paraît absolument nécessaire. Je suis évidemment défavorable à votre amendement j'en comprend le sens. Je voudrais vous dire également que l'accès aux classes préparatoires se fait sur sélection. Et que les élèves doit remplir les conditions requises. Des autres candidats, pour présenter pour se présenter au concours. Notamment les conditions diplôme. Très bien monsieur Vial. principes qui font que je suis là aujourd'hui, c'est la question de l'égalité des chances et de la méritocratie ces ces 2 valeurs qui qui ont fait que je je suis là aujourd'hui et il y a une différence quand même fondamental entre l'égalité des chances et ce qu'on essaye de faire passer pour de l'ouverture et de l'égalité, l'égalité des chances. C'est quoi ces données les toutes les les mêmes chances à tout le monde sur la ligne de départ, c'est-à-dire faire plus pour ceux qui ont moins de chances au départ de réussir leur donner les moyens de pouvoir réussir et ensuite une fois qu'ils sont sur la ligne de départ à égalité, c'est au mérite et à la compétence qu'il y arrive et c'est comme ça qu'on les détermine quand quand on on met en place des voies d'accès spécifique, c'est qu'on veut que tout le monde arrive. soi et gourou sur la ligne d'arrivée c'est plus de l'égalité des chances, c'est plus de la méritocratie. Si on a des des concours séparés. Si les compétences requises pour devenir magistrat ne sont pas les mêmes en fonction de de de votre niveau social ou de ce que faisaient vos parents. Alors je pense qu'on on on échappe un petit peu à ce que, à ce qu'ils font les principes fondateurs de la République et notamment la méritocratie l'égalité des chances qui doivent être au coeur d'une justice qui soit la même pour tous rendus par des des gens qui ont qui ont fait les mêmes études, qui ont les mêmes compétences pour rendre la justice et qu'on n'est pas une justice à 2 vitesses, donc à titre personnel je suis. Très favorable. Je reste très favorable à cet amendement. Je comprends les les. Des rapporteurs. Je suis par contre sur la question du principe et des arguments que vous y opposer pour maintenir ce cette cette. Cette sélection qui qui ressemble à de la discrimination positive. C'était en tout cas pas ma vision de de la République universelle. merci madame la présidente, circuler, je suis comme vous, très attaché aussi à l'égalité des chances ayant beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Dans ma ville du Havre. idem à la méritocratie. Je pense que c'est la récompense de ceux qui. S'investissent le plus dans leur parcours qui doit être reconnu et c'est justement le sens de ces de prépa talent les les le le le, l'objectif c'est de donner. Une chance à ceux qui ne ont pas naturellement parce que ils n'ont pas l'environnement. Ils n'ont pas les conditions pour préparer ce concours dans les mêmes conditions que les autres et on sait bien que malheureusement aujourd'hui l'accès à certaines filières reste difficile pour certains jeunes notamment issus des quartiers, d'autant que dans le dispositif prévu, ils sont soumis au même concours et aux mêmes conditions de crottes que tout le monde sauf qu'ils ont. Une prépa qui va les accompagner pour leur donner les mêmes chances de réussir ces concours. Et, et de même chance d'intégrer et dans l'intérêt de la justice parce qu'après ils auront une vision ils auront une ouverture. Ils auront une connaissance des problèmes qui sont liés à leur histoire, qui seront une plus-values, j'en suis convaincu, pour la magistrature. Merci je vais donc mettre aux voix cet amendement 35 qui a reçu un avis défavorable du gouvernement et un avis défavorable de la commission je vous remercierai de lever la main distinctement si j'ose dire pour le vote donc est pour. Qui est contre. Il n'est pas adopté. Le 23. Madame de La Gontrie. Il est défendu. Quel est l'avis de la commission sur ce 23 demandes de rapport défavorable. Monsieur le Ministre.

qui est contre qui s'abstient. Il est adopté. À l'article 12. On commence par le 22. 3 amendements identiques commenceront le. Dans trois amendements faisant l'objet d'une vision commune, toutes mes excuses. Le 22. Madame de La Gontrie est qu'il est défendu. Oui. Madame la présidente. Ça si vous allez défendent le 46. Merci madame la présidente. Cet amendement. Vise à permettre au gouvernement de prolonger la dérogation à l'application des quotas en matière de recrutements de magistrats actuellement le nombre de postes offerts aux candidats au concours professionnel est fixée par arrêté du garde des Sceaux, de la même manière que que pour les 3 premiers concours d'accès donc le texte proposé prévoit une dérogation à ces quotas pour les recrutements, qui auront lieu entre 2025 et 2028 dans le but donc de recruter 1500 magistrats d'ici 2027 et donc ces dispositions ne s'appliqueront pas s'appliqueront pas aux concours professionnel ouvert pour les années 2025 2006, 2007 et 2028 face à la possibilité d'une difficulté d'adaptation rapide des acteurs judiciaires aux nouvelles voies d'accès à la magistrature et au risque d'un système de quotas trop rigide. Nous, nous proposons donc avec cet amendement détendre la dérogation jusqu'à. 2031 pourquoi tout simplement pour assurer une transition plus souple vers les nouvelles modalités de recrutement en permettant aux acteurs judiciaires de mieux s'approprier les nouvelles voies d'accès à la magistrature. Bien. Le 57 n'est pas défendu donc madame Canayer le l'avis de la commission. Alors sur l'article l'amendement 22, pardon, c'est la durée du moratoire sur les côtés et les quotas professionnels au concours professionnel pardon. Donc votre amendement porte de 4 à deux ans, nous l'avons nous ramener à 3 ans pour rester dans le cadre qui est fixée pour la

par Madame Assassi. Alors on voit bien la volonté des avocats qu'on étende au maximum le moratoire pour qu'il puisse passer en nombre les concours et accéder à la profession de magistrats mais nous pensons que c'est pas une bonne solution, il faut offrir des chances à à tout le monde dans cette durée de trois ans, et pas au-delà. Avis défavorable. Monsieur le Ministre même. Même position, madame la présidente. Donc je me vois d'abord le 22 qui est pour. Qui est contre qui s'abstiennent n'est pas adopté 46 46 même votre j'imagine. Nous avons à 71 du gouvernement qui arrive maintenant. il est retiré par souci de cohérence. Madame la présidente. Idem pour le 85. Voilà, Neda et nous maintenant nous allons voter l'article 12 qui est pour. Qui est contre qui s'abstient. L'article 12 est adopté. Nous en avons terminé avec l'examen des articles de ce texte. Je vous rappelle que les explications de vote le vote auront lieu par scrutin public mardi 13 juin à 14h 30 la séance va être levé et la prochaine séance aura lieu le 12 juin, lundi 12 juin à 16h pour la proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public. La séance est levée. Merci à tous.